La séance est reprise. Alors j'ai informé le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française a été publiée. Cette candidature sera ratifié si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. La parole est à madame Marie-Noëlle Lienemann pour une mise au point, au sujet d'un vote. Oui madame la présidente, j'étais présente cet après-midi j'ai voté, j'ai vu le, le petit éclairage rouge et je suis notée comme n'ayant pas participé au vote. Je demande donc on rectifie et qu'on note que j'ai voté contre le scrutin lors du scrutin. 113. La parole est maintenant à monsieur Laurent Burgo a pour une mise au point également sujet. Merci madame le président. Je souhaite donc faire les mise au point suivante sur le scrutin public numéro 113. Mes collègues Jean-Noël Cardoux Laurence Garnier. Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir Anne Chain Larché souhaité voter pour. Merci à donné de vos mise au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique du scrutin concernés. nous reprenons la discussion de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants et dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'article. Nous avons 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 27 présentée par le gouvernement, Monsieur le Ministre. art, un amendement rédactionnel madame la présidente. Mais je peux effectivement précisé légèrement les dispositions prévues à paragraphe. 1 à trois auquel le gouvernement est favorable sur le fond permettront à la CPA de contrôler la bonne exécution des contrats par les assurances supprimons risque d'interprétation. À contrario des dispositions en vigueur. Oui madame la présidente. Il s'agit d'un amendement qui tend à éviter une dérive normative si l'article 7 précise effectivement que les prestataires de services remplissent bien leurs obligations contractuelles tout au long de la durée du contrat. Il me semble que dès lors que cela est convenu dans le contrat qui lie les parties. Il ne paraît pas nécessaire d'inscrire cela dans dans la loi c'est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette précision qui paraît superfétatoire. Merci l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Pour les deux. Merci beaucoup. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre sur le sept. Favorable. Quand je vais donc mettre aux voix l'amendement 27 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'article 7. Donc il a reçu un avis défavorable de la commission un avis favorable du gouvernement qui est pour.

Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je l'avais évoqué dans l'intervention général c'est sur l'utilité de l'est du que qu'à l'épargne retraite. Il est normal éventuellement complémentaires chacun puisse mettre de côté selon ses capacités financières durant sa vie au travail ou du 11, sa vie de rentier pour se garantir un niveau de retraite de vie tout à fait convenable. Et là. Notre groupe, pense au contraire que cette épargne massive l'encours de l'assurance-vie s'élevait à 1826 milliards en août 2022. Ce à quoi il faut ajouter les plans d'épargne action les plans et pas un gros traite les plans épargne logement et les plans. Que chacun pour lui-même ou les connaissais pas mais ils sont à la tête des gens, mais celui-là il est pas encore distribués. Vous m'avez compris cette masse d'épargne plus particulièrement les revenus qu'elle génère cotise aujourd'hui à 17 2 pour même lorsque sont exonérés d'impôt sur le revenu les rentes générées dans le même temps, on a le déficit du régime retraite qui pourrait atteindre à condition de financement équivalente. Je vais prendre les chiffres du conseil d'orientation des retraites. Plutôt que ceux d'un car les je pense le film Frank ultralibérale Molinari donc entre 7 5 et 10 milliards d'euros en 2027, ce qui fait 0 à 0,4,03, 0 4 point du PIB pour grimper entre 12, 5 milliards et 20 milliards à l'horizon 2032, 05 à 08 du point PIB donc les déficits seraient persistants sur les 25 prochaines années, même si la situation s'améliorera au long terme. Alors quand quand il est évoqué. Quand j'entends des fois des, des voix dissonantes qu'il faut travailler plus longtemps. Que nous rétorqueront que les travailleurs produisent des richesses qu'il convient de socialiser cet amendement s'inscrit donc dans le 7. Philosophie qui consiste à créer une contribution à 7 8 % éventuellement temporaire éventuellement temporaire le temps que l'ajustement démographique soit intervenu d'ici une quarantaine d'années sur les placements financiers. Donc voilà c'est un, un, un, un amendement responsable et je vous donne tout de suite le résultat s'il était voté le produit escompté serait de 650 millions d'euros. Merci. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapport. Qui a donné lieu ensuite à cette Pepel payer moins et gagner plus. Vous vous considérez qu'il faut taxer plus pour gagner moins. On est vraiment aux antipodes de l'objectif. En plus vous préempter pour le coup le débat dont nous avons souhaité et. C'est ce qui a été évoqué lors des débats en commission. Sur la question de la répartition capitalisation donc je je, vraiment je trouve que c'est un peu dommage, vous ne serait donc pas surpris de recevoir un avis défavorable.

Ce qui vous est proposé dans cet amendement ça amène. Un dixième du déficit du système de retraites avec une fiscalité totale. Toujours assez élevés puisqu'Helvète de 37 8 centimes par euro de plus va vu générés par ces placements. Donc franchement. Ça va pas épuisé toutes les sources de financement disponible voilà c'était son côté raisonnables. Merci. Alors donc je mets aux voix l'amendement 42 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre donc cet amendement et j'en ai parlé dans la discussion générale est un amendement de suppression de l'article 8. Je me réjouis de ne pas être le seul à le présenter, c'est-à-dire que. Au nom de la commission il soit également présenté je trouve que cela est sage. La proposition de loi qui nous est présentée. Elle vise à la protection des épargnants notamment. Dans un rapport qui est déséquilibré. Avec les assurances et les banques d'informations, de transparence, de concurrence et à remettre de l'équilibre et là cet article visait d'abord. Même si sa portée était très limité à proroger une incitation fiscale. Permettant d'investir vers un plan d'épargne retraite. C'est vrai que cette proposition de loi, un grand défaut, qui a dit Daniel Breuiller tout à l'heure c'est nous avoir empêché de manifester ou empêchés de manifester, plus d'un quart d'heure donc je me réjouis qu'il n'y ait pas d'articles qui favorise la retraite par capitalisation dans cette proposition de loi à partir du moment où nous en supprimerions l'article 8 dont la portée par ailleurs ne me semble pas essentielle. À la proposition de loi elles-mêmes donc j'en remercie. Par avance, Albéric de Montgolfier et Jean-François Husson et j'espère la la majorité du Sénat. Merci le 22 monsieur ça vole Denis. Merci madame la présidente, Rémy avait oublié de m'associer donc on on va faire la chaîne Rémi. Moi je m'associe à ce qu'a dit Daniel Breuiller, je m'associe à ce que tu as dit, et je m'associe à la suppression de l'article qui était c'est vrai par défaut. Mais une petite entrée à à la retraite par capitalisation de la suppression de cet article voilà merci. Merci. Si l'amendement 53 monsieur le rapporteur. Donc défendu ce qui me permet. De donner un avis favorable, comme on l'avait dit et je je veux juste rappeler, on va pas mélanger les genres. Albéric de Montgolfier à Amiens rappelé le travail de notre côté pour aboutir à ce texte remonte à 2020. Alors c'est vrai que. Convenez que nous n'avons pas choisi la date du jour de la manifestation aujourd'hui. Voilà au moins on a cet accord Pascale Daniel Rémy et les autres. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Avis favorable du gouvernement, alors même que c'est. Moi-même qui représente le le gouvernement ce soir au banques qui est conçu ce ce ce dispositif il y a 3 ans pour aller jusqu'en 2023 avec. La avec dans l'idée non pas de de fragiliser le système de retraite par répartition mais simplement tirant les les leçons de la loi pas qui avait harmoniser les produits d'épargne retraite. De faciliter le passage de l'épargne en assurance-vie utilisé par beaucoup de Français comme un produit de préparation à la retraite vers un produit qui a été conçu pour cela, c'est-à-dire le plan d'épargne retraite mais la la la phase d'acclimatation avec le nouveau PER et est sans doute désormais. Et donc il est, il est sans doute opportun. De mettre fin à ce dispositif désormais. Merci Monsieur le Ministre donc je mets aux voix ces trois amendements identiques à de 22 et 23 qui ont reçu donc un avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour.

Oui. Monsieur le rapporteur général tête pour vos agendas respectifs. L'intersyndicale. Je crois qu'il y a un mouvement qui est prévu le 7 février et puis après il y aura le 11 février dans c'est pour qu'on essaye de se coordonner quoi hein. je je vous remercie de le prendre avec sourire. Nous abordons à ce moment-là la question. Alors là ça va être un sujet aussi c'est l'opportunité pour la Caisse des dépôts d'administrer un fonds indiciel afin d'être distribués dans des plans épargne retraite. Le gouvernement aussi, mais je pense pas pour les mêmes raisons, mais je ne veux pas interpréter des propos qui n'ont pas été formulée. Mais je crois savoir que le gouvernement estime que le marché déjà suffisamment concurrentiel que la logique de chacun pour soi est un marché suffisamment porteur pour qu'un établissement public ne s'y intéresse. Mais vous me direz, Monsieur le Ministre, voilà d'abord si la proposition ne voulait s'intéresser à la façon dont la Caisse des dépôts pouvez contribuer encore davantage à la mobilisation de l'épargne populaire elle suggérerait d'augmenter le taux de centralisation faire en gros faire que pour un euros déposés sur un Livret A ou un Livret de développement durable et solidaire, ce ne soit plus de 60% qui puisse être centralisé mais 100% comme c'était le cas avant 1999. Le rapport de la Cour des comptes, tout le monde là en tête, forcément il date de 2010 donc ça nous fait revenir un peu en arrière ne dit pas autre chose en passant à 70% de centralisation 65% aujourd'hui, quitte à démanteler les fonds d'épargne qui sert à financer l'intérêt. J'ai général humain. Ce que je veux vous dire c'est que là on a un vrai sujet de l'autre côté. Est-ce que les fonds d'épargne sont forcément fortement sollicité par l'état non seulement pour le financement du logement social, mais aussi pour d'autres investissements d'intérêt général par exemple fin 2009, ceux-ci représentaient un encours de 11 milliards d'euros, soit 10% du total et concernaient des secteurs de plus en plus variés. Et des sujets qui nous importe aujourd'hui transport hôpital assainissement des eaux université. C'est donc pas à nos yeux une mission de la Caisse des dépôts, même lorsqu'elle se voit privés des ressources lui permettant d'assumer ses. Si collègue donc je vous dis ça parce qu'il y a un sujet NS c'est l'arrivée de BlackRock, madame la présidente. Oui on verra après. Tout à l'heure dans l'explication et maire. Si pour l'agenda hein. Merci beaucoup. Alors le 26 présenté par le gouvernement. Monsieur le rapporteur. Ce n'est pas tout de suite à vous-. Même si vous avez envie de répondre à Monsieur Savoldelli non vous allez attendre un petit peu. Merci madame la la présidente. C'est un amendement identique à celui de Monsieur. Savoldelli. Qui consiste à à dire que il n'est pas nécessaire que la Caisse des dépôts et consignations, créer un fonds de fonds indiciels car il existe d'ores et déjà des offres de marché d'ailleurs dans l'article 3 qui que vous avez adopté tout à l'heure, nous les mettons en visibilité dans les contrats d'assurance vie et dans les plans d'épargne retraite. C'est une très bonne chose, car ce sont des produits avec très peu de frais. Mais précisément, ce sont des des produits qui sont moins coûteux. À produire pour les les gestionnaires d'actifs. C'est la raison pour laquelle il t'y retrouve peu de frais, peu de coûts pour les pour les produire et il s'agit maintenant que ce marché se développe

De voir. La convergence d'un amendement défendu par Monsieur Savoldelli et par le gouvernement au moins. On va dire que le sujet. Donnent des points de vue divers et. Et ce qui me ce qui m'inquiète. Monsieur le Ministre, c'est l'argument que vous venez de donner, en disant, le marché est ouvert non. Le marché il est légèrement émergents il a principalement un opérateur et il y a besoin de l'ouvrir. Et l'idée de proposer, effectivement, un fonds de fonds indiciels côtés à Bakou. Et de proposer comme opérateur. La Caisse des dépôts, c'est qu'il faut avoir. Une taille suffisante et quelque part de pouvoir jouer de la concurrence. je suis encore surpris de voir. Nos collègues. Du groupe. Communiste défendre. Quasiment une situation aujourd'hui de monopole tenus par des opérateurs privés là ou de mon point de vue. Il y a besoin de mettre de la concurrence et effectivement l'objectif il doit être de favoriser l'épargne. Y compris au bénéfice de l'économie par les fonds de fonds indiciels côtés donc moins cher mais d'éviter. D'ouvrir les portes trop en grand à des opérateurs étrangers. Voilà notre objectif. Et voilà ce à quoi on invite les Français. Raison pour laquelle. Autant pour le goût. L'amendement du gouvernement que pour celui de notre collègue Savoldelli la vie les avis seront défavorables. Merci monsieur le rapporteur. Donc je vais mettre. Monsieur Savoldelli. mais. Merci madame la présidente sur le rapporteur général. Peut-être que je me suis mal expliqué. Moi ce que je vous disais. Et ce que je dis aussi au gouvernement, c'est que moi je ne suis pas en train de chercher à rivaliser avec un, un, un BlackRock à la française.

je vous cite, qu'un, je vais vous citer ceux qui mettent bas Croque la société américaine spécialiste de la gestion passive démocratisé c'est beau hein auprès du grand public, les fonds indiciels côtés qui reste l'apanage des institutionnels qui reste l'apanage des institutionnels. Qu'on doit pas sacrifier la rentabilité financière pour faire du bien à la planète. Vous voyez ce que c'est ça c'est ça que je dénonce moi donc il y a pas de collusion et etc, moi je défends nos institutions je défends l'investissement public l'intéressement public l'intérêt général. C'est ça la question alors que ils vous disent, non, non la rentabilité financière. Va plus importante que faire du bien à la planète CE donc c'est ça qu'on veut éviter, voilà peut-être un élément de de de clarification s'il en fallait un. Merci. Alors je mets aux voix donc les amendements, 23 et 26 identique amendements de suppression donc favorable du gouvernement défavorable de la commission qui est pour. Tu es contre. Ils ne sont pas adoptés je mets aux voix l'article 9 qui est pour. Qui est contraint qui s'abstient donc adopté. Tic le 10 c'est supprimé. Monsieur le rapporteur. Dans un monde idéal, j'avais même on nous avions même envisagé de le de, d'avoir un contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Ça sort un peu de sa mission traditionnelle et l'idée et se donner un peu de temps pour avoir. Un contrôle à priori, je dis bien à priori de cette information qui pourrait être au bénéfice des épargnants. Alors on est conscient du du délai. Donc c'est la raison pour laquelle, même en étant pas par principe très favorable au rapport. Nous sommes sur un sujet technique et donc on souhaite allonger le délai pour que le gouvernement nous fasse des propositions permettant d'avoir un contrôle efficace et a priori de cette information, en matière d'investissements défiscalisés d'Auxerre. L'amendement vise à porter de 6 mois à un an le délai pour la remise du rapport. Merci. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Le rapporteur a a évoqué la difficulté, c'est un avis défavorable en raison du délai. Merci donc je mets aux voix l'amendement 54 qui, qui est d'un amendement de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient donc adopté, je me vois l'article 11 qui est pour un contrat qui s'abstient donc adopté à l'article 12 l'amendement numéro 8 n'aime Paoli-Gagin. Oui madame le président. La nouvelle rédaction de cet article prévoit une obligation d'information pour tous les porteurs de projets qui ont bénéficié de services de financement participatif à compter du 1er janvier 2023. Cette disposition aura donc un effet rétroactif pour les plateformes de mise en relation qui auront commencé à collecter des fonds et et à. Ah les affecter à des projets d'investissement. Il est donc proposé de supprimer ce caractère rétroactif en repoussant d'un an, la date d'entrée en vigueur de la disposition pour permettre aux acteurs du secteur de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations. il y a pas de rétroactivité. On espère en tous les cas qu'ils ont quand même conserver la traçabilité. De l'ensemble des dons et des collectes donc avis défavorable pour ces trucs. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Même avis merci je mets donc aux voix l'amendement huit qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre un qui s'abstient. Il n'est donc pas adoptée, je mets aux voix l'article 12 qui est pour un contre qui s'abstient est adopté après l'article 12 l'amendement 15. N'est pas défendu.

Pardon, madame la présidente. Donc cet amendement vise à orienter les épargnants de contrats d'assurance-vie vers des investissements verts. On sait que les préoccupations environnementales sont une priorité aujourd'hui fondamental et qu'il y a besoin. De financement et donc en 2022 45 % des Français estiment qu'ils peuvent avoir un impact réel sur l'environnement et la société à travers leurs décisions de placement d'épargne donc. Les épargnants aussi des comportements citoyens durable je dirais et donc ces investissements verts sont un remède pour faire face à la crise écologique et aider à financer les investissements nécessaires. Je vous remercie. Tout à fait c'est un amendement donc qui vise aussi à orienter l'épargne essentiellement vers les investissements verts compte tenu que c'est une priorité aujourd'hui de l'action publique et donc il est nécessaire que le prendre des mesures permettant d'y aboutir. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Quand on commence comme ça, ça veut dire. Vous connaissez la suite. Donc. On partage l'objectif donc c'est voilà le mon néanmoins. Nous interrogeons sur le caractère opérationnel de cet amendement parce que. Peut-être que le gouvernement va pouvoir nous confirmer les chiffres d'après l'analyse de la Commission ignorait qu'un seul Label.

de des investissements en unités de compte qui soient des investissements verts donc voilà on partage objectif opérationnel. Pour cette raison, c'est plutôt une demande de retrait. Face une interrogation sur l'depuis. Au-delà de ça. Ça pose la question de la liberté de choix des investisseurs. C'est un autre question, est-ce qu'on doit imposer je jusque là actuellement il y a une choix une unité de compte euros faut-il au-delà pour l'instant, la commission n'y est pas favorable. Merci. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui madame la la présidente madame la présidente, monsieur le sénateur. Cette. Un avis qui sera le même que celui du du rapporteur simplement pour dire que. Dans le cadre de la loi pas ce qui a été fait c'est de d'introduire une obligation nouvelle, celle pour les distributeurs de contrats d'assurance vie ou pour les, les, les compagnies d'assurance, de présenter au moins une option sociale une option environnemental et ça a permis de faire en sorte que désormais tous les catalogues d'unités de compte. Qui sont présentés au au client. ce ce type d'offre. Mais là vous êtes effectivement particulièrement ambitieux en demandant ce les les certains des catalogues d'unités de compte sont quand même très étendu. Est ce que vous proposez avec votre amendement c'est que. Vous va soit 25% soit 50%. Reflète les les les le Label Green fine ce qui ce qui effectivement peut être trop ambition à ce stade, même s'il n'est pas exclu qu'on y parvienne. Dans les années qui viennent. Merci monsieur K. Oui merci madame la présidente. Alors effectivement je pense qu'il faut être ambitieux dans la vie. Parce qu'aujourd'hui il y a des objectifs. Ambitieux en termes de transition énergétique entre terme de transition écologique. Et donc il est nécessaire leur plus avancer là-dessus. C'est l'objet de ces amendements. Merci alors je mets aux voix donc l'amendement 13 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

Oui madame le président. Cet article en fait, instaure un pouvoir d'astreinte au bénéfice de l'AMF qui lui donnerait davantage d'effectivité. En terme de pouvoir d'injonction. Il renforce cependant également le caractère unilatéral de la décision qui font que l'injonction en assortissant cette décision d'un effet de sanctions immédiates. Mon amendement. À défaut d'encadrer le pouvoir d'astreinte précise ainsi que le collège de l'AMF et tenus de mener une procédure contradictoire avant de déterminer une injonction. Merci beaucoup. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur.

Là on n'est pas une sanction dans une astreinte avant de projeter. Avant de prononcer. Une astreinte donc est ce qu'il faut-il aller jusqu'à une mesure contradictoire parce que maman peut nous peut nous éclairer sur ce point en l'état actuel, ça nous paraît. En tous les cas, couvert au moins partiellement par le l'article L 621 14 du code monétaire et financier. Merci. Donc l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présente pour répondre. Au rapporteur, c'est déjà le cas dans le cadre du collège et donc. L'avis du gouvernement, est le même que celui du rapport. Merci donc je mets aux voix l'amendement numéro 9 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre contraint qui s'abstient n'est pas adopté l'amendement 55 de la commission. Monsieur le rapporteur. Coordination pour l'application en outre-mer. Merci Monsieur le Ministre même avis enfin favorable donc je mets aux voix l'amendement 55 de la commission qui a reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient donc adopté. Je me vois l'article 13 qui pour contre, il est adopté. Je me vois l'article 14. Ce même votre. Article 15 même votre. L'article 16 même votre l'article 17 même vote. Et un article additionnel après l'article 17. Monsieur le Ministre, l'amendement 25. Oui madame la présidente. Avec cet amendement, nous remet Dion à à l'imprécision de l'article L 621 14 du du Code monétaire et financier sur les modalités de recouvrement du montant des astreintes prononcées par le président de la cour d'appel de Paris sur du président de l'Autorité des marchés financiers. L'impossibilité de recouvrer ses sommes diminue la portée du pouvoir d'injonction de l'AMF. Il est toutefois nécessaire d'assurer l'effectivité des décisions du superviseur pour préserver sa crédibilité et assurer la pleine intégrité des marchés. Merci la vie, la commission monsieur le rapporteur. Favorable, favorable. Merci je vais donc mettre aux voix l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission le 25 qui pour ces contre qui s'abstient. Il est donc adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Je vais donner la parole à monsieur Savoldelli pour explication de vote. C'est en effet madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors je ne vais pas vous parler du 49.3 je ne vais pas parlé du 47 hein, je vais vous parler de l'Arctique. 45. Des amendements qu'on avait proposé qu'on était hors sujet. Voyez avoir c'est simple. Plafonner les frais de tenue de compte à 12 euros par an hors sujet. Suppression des frais d'incident pour 4, 1 millions de clients en situation de fragilité financière allocataires du RSA des APL de l'allocation adulte handicapé aux étudiants boursiers hors sujet. Suppression des frais bancaires pour les saisies administratives attire des tendeurs c'est-à-dire pour des personnes qui auraient des dettes fiscales ou des arrêtés de factures de cantine ou d'hôpital par exemple. Hors sujet pareil. Enfin, plafonner les frais d'incidence pour les comptes des professionnels des auto-entrepreneurs des travailleurs indépendants. Allez on ne va pas faire de, on ne va pas les citer Hubert Deliveroo et toute la bande qui, qui organise les plateformes numériques de de travail. Je vous le dis par exemple Hubert le salaire mensuel c'est 1617 euros et ils font 45 3h par semaine en moyenne. Et bien entendu c'est pas 35 40 là. Et ben ces travailleurs et travailleuses qui roule pas sur l'or, c'est le moment de le dire avec la ponction de l'application 25% il devrait subir la ponction des banques via des commissions d'intervention, tout ça pour vous dire à travers ces ces amendements qui ont été frappés par l'45, que le projet de loi qui est là certes protège les épargnants en partie d'ailleurs vous avez vu qu'on a eu des votes positifs et constructifs. Mais franchement il y a un problème c'est que. C'est c'est qu'on fait rien sur l'épargne financiarisé on la cible pas on l'oriente pas voilà c'est c'est à l'aveugle. Donc c'est de la valeur pour la valeur. Alors je dis pas il ne faut pas faire de la valeur pour la valeur. On ne peut pas faire que de la valeur pour de la valeur. Il y a l'économie à l'emploi, il y a des défis climatiques les défis sociaux qui sont devant nous. Donc voilà c'est pour expliquer comme je l'ai dit dans l'intervention générale que nous voterons contre cette proposition, merci. Merci. Alors je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient et donc adopté. La on ne va pas suspendre va continuer tout de suite. Si chacun peut prendre sa place. Rapidement. Merci beaucoup. l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti Garde des Sceaux, ministre de la justice. Monsieur le ministre, c'est à vous.

madame la présidente. Monsieur le Ministre, cher Olivier. Monsieur le président de la commission des lois. Madame, monsieur les rapporteurs mesdames et messieurs les sénateurs. La proposition de loi que vous examinez aujourd'hui. Dans le temps réservé au groupe RDPI. Vise à apporter une. Réponse indispensable à des situations. Individuelles auxquelles je suis particulièrement sensible. Et qui concernent la vie quotidienne. De femmes et d'hommes que nous essayons chacun à notre niveau d'améliorer chaque jour. Je vous ainsi d'abord remercier. Le président Patriat et ses collègues qui ont permis de poursuivre les travaux. De l'Assemblée, au Sénat dans des délais extrêmement brefs. Au cours des derniers mois, nous avons été. Nombreux. À être saisie par. Des petits propriétaires qui ayant. Économisé toute leur vie pour acquérir un bien. Se retrouvent dans l'impossibilité de récupérer le fruit de leur travail et de leurs économies. Je pense en particulier. À l'exemple. Frappant. D'une vieille dame vivant dans un Epad. Qui s'est retrouvé dans l'incapacité de reprendre possession de son appartement. Squatté. Qu'elle souhaitait vendre pour payer les mensualités de son Nepad et assurer ainsi sa fin de vie. Impossible de récupérer son bien. Car l'appartement était occupé. De façon illégale. Cette situation évidemment est intolérable et porte gravement atteinte. À notre pacte social et républicain. Lequel veut que les citoyens s'en remettre aux autorités. Tout simplement pour faire respecter la loi. Il est inacceptable qu'une dame âgée. Angoisse à l'idée de ne plus pouvoir payer ses traites parce qu'elle ne peut pas récupérer un bien acquis. Après des années de labeur. Je le dis tout Net. La lutte contre les squats et nécessaire et la priorité de ce gouvernement et en particulier de mon ministère. Dans cette lutte. Force doit rester à la loi. Laquelle doit protéger les honnêtes gens. Je veux d'abord rappeler. Je dois d'abord rappeler. Que la protection du droit de propriété figurent au nombre des droits de l'homme consacrés par la déclaration de 1789. Toutefois, ce n'est pas le droit de propriété que protège aujourd'hui le délit de l'article 226 IV du code pénal. Mais le domicile comme émanation. Du droit au respect de la vie privée, lequel est constitutionnellement et conventionnellement garantie. C'est l'objet du délit de violation de domicile. Depuis 2015, l'article 226 tiré IV distingue expressément 2 infractions. Dont celle de maintien dans le domicile d'autrui qui présente la particularité d'être une infraction continue et non une infraction instantanée comme l'est l'introduction dans le domicile d'autrui. Cette particularité fait que les forces de l'ordre peuvent tout au long de l'occupation intervenir et interpeller les squatteurs, quel que soit le délai écoulé 48 heures ou plus, depuis leur introduction dans le domicile. Cette infraction est donc un outil juridique efficace et puissant pour faire cesser les situations de squat caractérisé, j'insiste sur ce fait, car il est trop souvent cité dans la presse des cas de Français partis en vacances, qui ne peuvent pas récupérer leur domicile car plus de 48 heures se serait écoulé. Concernant spécifiquement ce délit de violation de domicile. La proposition de loi apporte 2 améliorations. En 1er lieu. La ligne les peines sur celles encourues par le propriétaire qui par exemple expulse le squatters qui occupent son domicile. Un tel alignement dans l'échelle des peines me semble absolument nécessaire et permettra de répondre à une situation que nous pouvons qualifié de totalement injuste. En second lieu elle clarifie la notion de domicile en précisant qu'elle recouvre tout local d'habitation contenant des biens meubles qu'une personne il habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non cette clarification est bienvenue puisqu'elle permettra, je l'espère, de faire cesser les fausses informations sur l'étendue de ce délit. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment certains médias le squat d'une résidence secondaire. Hé bien constitutifs du délit de violation de domicile, comme je l'ai déjà expliqué, s'agissant d'une infraction continue l'intervention des forces de police pour faire cesser cette situation est possible à tout moment. Ça va s'arranger. C'est l'objet de ce texte, monsieur le sénateur. La proposition de loi entend aller au-delà de la protection du domicile en protégeant également la propriété en tant que telle, une telle évolution est indispensable pour mettre fin aux situations injustes que j'évoquais précédemment. Il nous faut toutefois nous assurer que ces infractions sont suffisamment ciblée et ne vont pas au delà de ce qui est nécessaire. Il ne s'agit ainsi pas de faire primer le droit de propriété sur toute autre droit social, mais de répondre de manière proportionnée et adaptée à des situations individuelles. Profondément injuste. À cet égard, je tiens à souligner l'important travail des commissions des lois et des affaires économiques dont je veux ici saluer les rapporteurs, le sénateur Richard et la sénatrice Estrosi Sassone engagé de longue date sur ces sujets. Leurs travaux ont permis de resserrer le Champ du délit d'introduction ou de maintien dans un local autre que le domicile. Les travaux de vos de commission. Ont permis d'aboutir à un texte qui me semble satisfaisant à plusieurs égards. Tout d'abord vos travaux ont permis de préciser le Champ de la répression aux seuls actes frauduleux en prévoyant s'agissant des locaux, autre que le domicile que l'introduction à l'aide de manoeuvres, menaces voies de fait ou contrainte ou le maintien après une telle introduction sont réprimées. Cette restriction du Champ de l'infraction permet de répondre aux inquiétudes exprimées par certains et aux réserves que j'avais émises lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale en excluant de la répression, les locataires défaillants qui ne font l'objet d'aucune mesure. D'expulsion nos débats. n'en point douter permettront de parfaire plus avant le texte, en précisant le terme local à usage économique qui ne correspond à à aucune notion connue dans notre droit. Il me semble également opportun de réserver la protection aux seul locaux effectivement. Exploiter. Dans la lutte contre les squats. Votre commission a également procédé à une gradation dans l'échelle des peines qui me semble tout à fait bienvenue. Sur l'aspect pénal du texte. Il me semble donc que les travaux de vos commissions ont permis d'aboutir. un équilibre entre la défense de la propriété immobilière, qui concerne aussi les petits propriétaires. Et le droit au logement dans le respect de nos principes constitutionnels. En complément des outils ou fait ou offert pardon. Par notre procédure pénale. Nous disposons de devoir pour expulser le squatteur du logement d'autrui une voie civile. Et une voie administrative la voie civile permet de saisir le juge des référés. Celui-ci lorsqu'ils. Constatent l'existence d'un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire l'occupation du bien peut ordonner les mesures conservatoires qui s'impose, dont l'expulsion. Le délai moyen de cette procédure, et de 5 mois. Nous disposons également depuis la loi Dalo. D'une procédure administrative. D'évacuation forcée. Son article 38. Permettent aux préfets lorsqu'une plainte a été déposée pour violation de domicile. D'ordonner l'évacuation des squatters sans attendre qu'une décision judiciaire était. Rendu. À la suite de la loi ASAP. Qui est venue compléter la loi Dalo. Nous avons pris l'initiative avec mes collègues des ministères de l'Intérieur et du logement d'adresser le 22 janvier 2021 une instruction aux préfets pour détailler la mise en oeuvre de cette procédure et leur enjoindre d'assurer la rapidité de son exécution. Plus que jamais, l'exécutif et donc mobilisés pour lutter contre les squats. Tout en en conservant l'esprit de la proposition de loi du président Kasbarian votre commission a recentré son application aux squatters. Je m'en félicite car la procédure de l'article 38 n'est pas adaptée à l'évacuation des autres types d'occupants, locataires concubins. En raison de son caractère expéditif et non contradictoires. Je pense notamment à la situation dans laquelle se seraient retrouvés une femme victime de violences conjugales dont le compagnon violent serait partis sur ordre de la justice mais qui aurait quand même pu exiger du préfet une évacuation forcée de sa victime. La nouvelle rédaction de l'article 2 de la proposition de loi a également clarifié l'extension du périmètre de cette procédure, elle sera mobilisable pour la libération des domiciles mais également des logements vacants. La question des expulsions pour impayés de loyer. Et quant à elle bien distincte de celle du squat. Il faut garder à l'esprit que notre droit civil. Protège les locataires qui cesse temporairement de payer leur loyer. La difficulté à régler une échéance de loyer. En raison d'un accident de la vie ou de facture imprévue ne doit pas compromettre définitivement le logement familial, le texte adopté en commission rétabli sur ce point le pouvoir du juge d'accorder d'office des délais avant

La condition ajouté par votre commission à l'octroi de délais par le juge s'inscrit, me semble-t-il dans l'équilibre que nous recherchons entre droit au logement et droits de propriété. Pour autant, cet équilibre est fragile car on sait que 40% des locataires en impayés ne se présente pas à l'audience et ignorent leur droit de demander des délais dès lors que l'expulsion est ordonné, le juge peut encore octroyer de façon exceptionnelle des délais supplémentaires afin de permettre à des familles en situation de précarité de se reloger dans des conditions dignes. Le droit civil fait également obstacle aux expulsions durant la trêve hivernale. C'est là un acquis non négligeable. J'insiste sur ce point car la loi Veil ainsi à répondre à des situations individuelles qui peuvent se révéler dramatiques, il n'apparaît pas souhaitable. Que la légitime lutte contre les abus de locataires de mauvaise foi conduisent à modifier ces équilibres. La proposition de loi prévoit la réduction de certains de ses délais de procédures afin d'accélérer le traitement de ces affaires. Si j'étais favorable à la réduction de ces délais à deux mois. Je considère trop court et difficile à calculer, celui de six semaines voté en commission. Ainsi, s'agissant des propriétaires. Il est important de sécuriser leur situation face à des situations si. À des occupations illicites de leurs biens et donc. De les décharger dans certaines circonstances, de leur responsabilité, c'est l'objet de l'article 2 bis de la proposition de loi. Cependant les décharger totalement de leur obligation d'entretenir leurs biens nuirait de manière injustifiée au tiers subissant un dommage c'est tiers doivent pouvoir être indemnisé sans supporter les conséquences d'une occupation illicite. Une nécessaire adaptation de ce texte devra être envisagée. C'est le sens de certains amendements dont un à l'initiative du gouvernement qui seront proposées à votre vote tout à l'heure. Dans la lutte contre les squats et la préservation du droit de la propriété. Ce texte est une nouvelle étape intéressante, faisons en sorte tous ensemble qu'il apporte des solutions efficaces, concrètes, dans le respect de nos grands principes constitutionnels. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à monsieur Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, chez Éric. Monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur de la commission des lois. Madame le rapporteur de la commission des affaires. Faire économique mesdames et messieurs les sénateurs. Vous avez aujourd'hui à examiner un texte qui traite de situations humaines souvent complexe. Des situations humaines qu'en tant qu'élu nous connaissons vous connaissez. De cette expérience d'élu. Vous savez la différence entre les situations inacceptables de squats et les situations relatives à des impayés de loyers. Fort de ses expériences. Vous examiner ce soir un texte équilibré qui ne confond pas ces deux cas dissemblables. Vous examiner un texte équilibré et même améliorée. Je salue à ce titre à mon tour tout particulièrement le travail des rapporteurs qui ont été attentif aux inquiétudes que pouvait susciter ce texte sans renoncer à l'ambition initiale d'apporter des réponses à certains cas insupportable. J'espère que notre discussion permettra de continuer à mieux distinguer la sieste situation du squatters qui doit être sanctionné à la mesure de sa faute de celle du locataire défaillant qui doit pouvoir être accompagnées lorsqu'il est de bonne foi. En effet. S'il est nécessaire de rééquilibrer de sécuriser les rapports locatifs. Et d'entendre les problématiques des propriétaires. Il faut aussi répondre aux locataires qui rencontrent des difficultés en les accompagnant le plus en amont possible. Il est donc primordial de bien distinguer le squatteur qui rentrent illégalement dans un domicile du locataire qui rencontrent des difficultés pour payer son loyer. Grâce à un amendement du président Patriat que je remercie et à travers lui l'ensemble du groupe RDPI pour les échanges fructueux que nous avons eu il y a par exemple une graduation entre la peine encourue pour le squat de domicile et celle prévue pour le squat de locaux économique. Et j'espère que l'examen permettra de préciser la notion comme ça vient d'être rappelé de locaux économique, de sorte que demain un squatteur soit sanctionné. Si l'équipe un local exploité et que toutes les entreprises dont les bureaux sont vacants utiliseront le beau dispositif d'occupation temporaire que nous avons pérennisé à l'Assemblée et que vous avez sécurisé en commission. En utilisant un dispositif légèrement différent de la version initiale. Le texte maintient et renforce les sanctions et j'en suis très heureux pour bien connaître ce problème dans ma ville contre les marchands de sommeil. Ce qui indument organise des squats en faisant croire qu'ils sont propriétaires de logements en toute illégalité et au détriment des plus faibles. C'est inacceptable et le gouvernement est pleinement mobilisée contre ce phénomène. Cela s'inscrit d'ailleurs dans la lutte du gouvernement contre l'habitat indigne, dont les procédures ont été renforcé et simplifié par la loi Elan adopté lors de la précédente législature. Concernant le traitement des locataires en impayés de loyers. Je me satisfait vraiment que la commission est maintenu les pouvoirs d'office du juge pour définir un plan d'apurement de la dette locative et vérifier les éléments constitutifs de cette dette. Le gouvernement l'avait déjà soutenu à l'Assemblée nationale dans une version un peu plus large pour tous les locataires de bonne foi. La navette pourra permettre d'évoquer cette disposition mais je veux dire ici, tout le soutien du gouvernement à cette évolution positive pour les locataires et pour les bailleurs dont l'intérêt que le locataire paie rapidement son loyer et rembourse ses dettes des après l'audience. La proposition de loi vise aussi à accélérer les procédures. À propos du délai légal entre le commandement de payer et l'assignation en justice le gouvernement salue le travail de la commission de passer ce délai de un mois à six semaines. Toutefois, comme vient de le rappeler le garde des Sceaux nous souhaitons le maintenir à deux mois à la fois pour éviter l'engorgement des tribunaux. Et pour plus de lisibilité car les paiements des loyers sont bien sûr vous le savez, la plupart du temps mensuelle. Enfin, je tiens à souligner le travail de la commission des affaires économiques qui a permis d'instituer des dispositions nouvelles afin de permettre un meilleur accompagnement social des locataires défaillants en renforçant les pouvoirs et l'information des Capes.

Ou encore des pouvoirs renforcés pour maintenir les APL ou demander le versement des aides directement au bailleur. En parallèle de ce texte. Je veux rappeler ici que le gouvernement continue à être prenne pleinement mobilisés pour prévenir les expulsions locatives. Je souhaite d'ailleurs que la prévention constitue un axe du plan logement d'abord de. Des outils de prévention sont déjà déployés dans le cadre du plan interministériel de prévention des expulsions avec par exemple, vous le savez le déploiement d'équipes mobiles. Plus de 70 équivalents temps plein, financés par l'État. Les fonds de solidarité pour le logement accompagne également les locataires en particulier dans la période actuelle des hausses de charges. Au-delà des bouclier tarifaire et de l'accompagnement mises en place par le gouvernement, notamment avec le chèque énergie. C'est aussi pour cela que je crois très important de conserver tous les efforts faits dans la prévention des expulsions locatives. Il faut laisser le temps du travail social. Il faut laisser au juge le pouvoir d'analyser chaque situation d'être au plus proche des réalités difficiles d'une expulsion qui est toujours un échec. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Ce texte que vous avez à examiner est équilibré. L'équilibre apaise le marché évite des cautions toujours plus importante des assurances toujours plus cher des cautions locatives porté par des garants qui sont discriminante et inégalitaire. Mais il ne doit pas se faire en ignorant les situations humaines, des locataires les ruptures et les heures. J'ai confiance dans l'esprit de discernement du Sénat pour préserver l'équilibre de ce texte auquel le gouvernement donnera un avis favorable. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à monsieur André Reichardt pour. Rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes, chers collègues. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues. L'examen de la proposition de loi visant à protéger les jaunes, les logements contre l'occupation illicite nous donne l'occasion de revenir sur 2 sujets auxquelles le Sénat et depuis longtemps attentif. La lutte contre le squat et la sécurisation des rapports locatifs. Il y a 2 ans à quelques jours près, le Sénat débattait sur le rapport d'Henri, le roi de la proposition de loi de notre collègue Dominique Estrosi Sassone visant à mieux protéger la propriété privée contre le squat. Plusieurs dispositions que le Sénat avait alors adopté sont reprises dans le texte qui nous faisons tout ce Nous sommes nombreux à regretter que le gouvernement n'ait pas été plutôt monsieur. Garde des Sceaux à l'écoute des propositions du Sénat, ce qui nous aurait permis de gagner du temps, un temps précieux pour lutter contre le phénomène du squat qui affecte vous l'avez dit tout à l'heure régulièrement des petits des petits propriétaires qui découvrent par exemple en rentrant de vacances, vous l'avez dit aussi que leur résidence principale est occupée. La première partie du texte qui nous est soumis, vise à prévenir et à réprimer plus efficacement le squat. La commission des lois, ainsi que la commission des affaires économiques, saisie pour avis ont veillé à mieux distinguer la situation du squatteur de celle du locataire défaillant dont le mail dont le bail a été résilié, mais qui s'était introduit régulièrement dans les locaux. Le texte comporte d'abord une série de dispositions en matière pénale. Certaines avaient d'ailleurs déjà été adoptés par le Sénat en janvier 2021, rapporteure de la commission des affaires écho je pense par exemple à la Redoute l'alourdissement de la peine encourue encourues en cas de squat d'un domicile, ainsi qu'à la création d'une infraction pour punir d'une amende la propagande ou la publicité en faveur de méthodes visant à inciter ou faciliter le squat. Vous savez comme moi que l'on peut trouver sur Internet de véritables guides du squat. Qui donne des conseils sur la manière de s'introduire illégalement dans un logement et d'échapper à l'expulsion. C'est ce type de pratiques qui seraient désormais pénalisée. Actuellement, vous le savez, le code pénal sanctionne seulement le squat du domicile sur le fondement du droit à la protection de la vie privée. Afin de garantir le droit de priorité de propriété qui est aussi un principe fondamental dans notre République. Le texte résultant des travaux de la commission crée une nouvelle infraction pour sanctionner le squat de locaux qui ne constitue pas un domicile. Le texte prévoit également une peine pour les locataires du parc privé qui se maintiennent sans droit dans leur, dans leur logement alors qu'ils sont sous le coup d'une décision définitive d'expulsion et qu'ils ont épuisé tous les délais accordés par le juge. Je sais que cette dernière mesure est contestée. Mais je pense qu'elle peut envoyer un signal à l'encontre de certains locataires d'une particulière. Mauvaise foi et je sais pouvoir faire confiance à la justice pour l'appliquer avec discernement. Le texte revient ensuite sur la procédure d'évacuation forcée des squatters sous l'égide du préfet prévue à l'article 38 de la loi instituant le droit au logement opposable, dite loi Dalo. Cette procédure permet à celui dont le domicile est squattée de saisir le préfet afin qu'ils mettent en demeure dans un délai de 48 heures le squatteur de quitter les lieux. Cette procédure dérogatoire qui ne fait pas intervenir une décision de justice a été utilisé, nous dit-on, environ 170 fois au cours de l'année écoulée. Sur ce point. La commission a décidé de rein réintroduire des décisions que nous avions adopté il y a 2 ans mais qui n'avait pas été reprise. L'objectif est d'abord d'élargir le Champ d'application de cette procédure à l'hypothèse du squat de logements qui ne constitue pas un domicile, ce qui est cohérent avec les mesures envisagées en matière pénale ainsi à logement qui est squattée alors qu'il est vide entre 2 locations par exemple pourraient être libérés rapidement également. Il s'agit ensuite de prévoir que la préfecture sollicite l'administration fiscale afin d'établir les droits du propriétaire dans le bien et squattée lorsque bien entendu l'occupation illicite, l'empêche d'accéder aux documents lui permettant de prouver que le bien lui appartient. Ces documents se trouvant dans le. Logement squatté. Enfin le texte ramène de 48 à 24h le délai prévu pour procéder à la mise en demeure. Dans un autre registre, mes chers collègues, la commission a approuvé le régime dérogatoire de responsabilité civile applicable aux propriétaires d'un logement occupé sans droit ni titre en cas de demain de dommages résultant d'un défaut d'entretien en prévoyant cependant une exception pour les marchands de sommeil. Il ne nous paraît en effet pas normal qu'un propriétaire qui ne peut plus accéder à son bien soit condamné en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien. La commission s'est également prononcé en faveur de la pérennisation du dispositif expérimental. Créé en 2009, de mise à disposition temporaire de locaux vacants. Même si nous regrettons que messieurs les Ministres l'évaluation que le gouvernement devait produire n'ait jamais été réalisé. Les auditions auxquelles nous avons procédé avec. Madame Dominique Estrosi Sassone monstre que ce dispositif joue un rôle utile. 10.000 personnes et ce n'est pas rien en ont bénéficié jusqu'ici et qu'il contribue indirectement à la lutte contre le squat, en favorisant l'utilisation de locaux provisoirement inoccupés. La seconde partie du texte vise à sécuriser les rapports locatifs en améliorant la procédure contentieuse. Le contentieux locatif est aujourd'hui soumis à une procédure complexe qui durent parfois des années dont les objectifs premiers sont dans l'intérêt du propriétaire, comme du locataire, le maintien des des rapports locatifs et l'apurement de la dette. L'expulsion pour nous reste la solution de dernier recours, a fortiori si le locataire en difficulté naturellement et de bonne foi. Il s'agit d'un contentieux de masse qui occasionne chaque année la délivrance, tenez-vous bien, de 500.000 commandement de payer et 150.000 assignations en justice pour 70.000 décisions d'expulsions ferme dont 16.000 nécessite le concours de la force publique. La réforme contribuera, nous l'espérons. A redonner confiance aux propriétaires qui hésitent parfois à mettre leurs biens en location, de peur de ne pas pouvoir le récupérer en cas d'impayés de loyers ce rétablissement de la confiance est indispensable, alors que des millions de nos concitoyens sont mal logées. Les locataires n'ont pas non plus intérêt à ce que les procédures judiciaires s'éternisent. S'ils veulent éviter d'accumuler une dette locative qu'ils ne parviendront alors là certainement plus à rembourser. Dans un souci de sécurité juridique. Il est d'abord proposé de généraliser les clauses résolutoire de plein droit dans les baux locatifs. En cas d'inexécution du contrat. La présence d'une clause résolutoire permettra aux propriétaires de saisir rapidement le juge pour qui l'on constate la résiliation. L'Assemblée nationale avait par ailleurs souhaité réduire certains délais et elle avait subordonné certaines facultés reconnu au juge à une demande expresse du locataire dans le but affiché afficher de le responsabiliser. La commission des lois à retoucher ses dispositions en effet beaucoup de locataires connaissent mal leurs droits et ne sont pas familiers de la procédure. On nous l'a dit souvent lors des auditions, il nous a paru important que le juge puisse de sa propre initiative leur accorder un délai avant la résiliation du bail pour qu'ils puissent d'une part vérifier les éléments constitutifs de la dette locative et d'autre part, s'assurer de la décence du logement. Nous avons également décidé de porter d'un mois, six semaines, le délai entre le commandement de payer l'assignation devant le tribunal car ce délai est souvent mise à profit pour régler à l'amiable les litiges les litiges locatifs dans plus des 2 tiers des cas. Je reviendrai tout à l'heure sur des amendements allant en sens inverse pour expliquer pourquoi ces six semaines sur proposition de la commission des affaires économiques. Nous avons enfin introduit dans le texte. Un nouveau chapitre destiné là encore à améliorer l'accompagnement social des locataires en difficulté, notamment en renforçant les prérogatives des commissions des coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Les CAPEX qui existe dans chaque département, il est important que ces commissions puissent travailler plus en amont. Si l'on veut que leurs efforts de prévention des expulsions produisent vraiment leurs effets Dominique Estrosi Sassone aura l'occasion de revenir plus en détail sur ces mesures. Dans quelques instants. Au total, mes chers collègues. Messieurs les Ministres, madame la présidente, vous voyez nous nous sommes efforcés d'aboutir à un texte qui réponde aux attentes des propriétaires sans fragiliser la position des locataires qui peuvent connaître un accident de la vie ou qui ont alors besoin d'être soutenus. Nous avons cherché à concilier le respect de la propriété privée et le droit au logement qui est un objectif de valeur constitutionnelle. Pour ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à soutenir le texte qui a été qualifié tout à l'heure par les ministres d'équilibrer et que j'appelle moi aussi équilibré telle qu'il est issu des travaux de notre commission je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques pour cinq minutes. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre commission des affaires économiques s'est saisie pour avis de l'intégralité du texte de cette proposition de loi car en même temps que les dispositions de droit pénal et de procédure civile a d'exécution. Elle contient des dispositions qui auront un impact sur la politique du logement, la lutte contre les squats. Le règlement des impayés de loyers et in fine et la prévention des expulsions. Car si d'un côté force doit rester à la loi. Face à la violence des squatters et des occupations illicites le domicile et la propriété devant être mieux respectée. De l'autre côté, cela ne peut et ne doit pas conduire à mettre à la rue des familles Dick Tim d'accidents de la vie qui ont besoin d'un accompagnement précoce et adaptée. Avec André Reichardt que je remercie et avec qui nous avons travaillé de manière très constructive. C'est cet équilibre que nous avons voulu trouver on étant plus strictes avec les squatteurs et les locataires de mauvaise foi. Tout en assurant une meilleure prévention des expulsions, sans en faire porter le poids sur les propriétaires. Le squat. Vous l'avez dit monsieur le garde des Sceaux est un véritable viol de l'intimité et la Commission veut qu'il soit réprimer sans faiblesse. Au delà des squatters. Nous devons nous attaquer aux réseaux organisés qui promeuvent et organise le squat y compris en utilisant et en abusant de la bonne foi de certains locataires. Il faut protéger non seulement les domiciles mais aussi les futurs domicile une personne réalisant son rêve d'accéder à la propriété et qui vient d'acheter son logement ou un ménage qui se voit enfin attribuer un logement social peuvent être privés de la jouissance de leur habitation par des squatters. Ils méritent eux aussi d'être protégées. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Je crois aussi qu'il nous faut sortir d'une vision dans laquelle on excuse le saut le squat soit vis-à-vis de supposés riches propriétaires. Soit en raison de la crise du logement. La réalité c'est qu'à Paris, environ un quart des victimes de squats sont des locataires. La réalité c'est que 2 tiers des propriétaires n'qu'un bien en location bien souvent pour compléter une retraite arrêtons également d'excuser l'occupation illégale de locaux vacants alors même qu'existent à travers le logement temporaire que nous allons pérenniser et sécuriser dans ce texte, un dispositif légal permettant à des entreprises agréées ou à des associations d'insertion, d'organiser un hébergement à destination des personnes en mobilité ou en grande fragilité. Arrêtons enfin de faire porter aux propriétaires le poids d'une politique défaillante du logement. Car si les constructions et les possibilités d'attribution ne sont pas assez nombreuses. Ce n'est pas de la faute des propriétaires mais plutôt de celle du gouvernement sur le sujet du squad d'ailleurs que de temps perdu. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, le Sénat a voté la proposition de loi que j'avais présenté pour mieux le réprimer plusieurs problèmes seraient d'ores et déjà résolu si elle avait été votée à l'Assemblée nationale alors que plusieurs de ses dispositions sont reprises dans ce nouveau texte concernant l'accélération des procédures d'impayés d'expulsion nous approuvons l'objectif général car la longueur des procédures décourage les propriétaires d'investir et de proposer des logements à la location de longue durée pour préférer des meublés de tourisme cette protection exagéré se retourne donc contre les locataires et se traduit par une pénurie de logements à louer. Pour autant, nous avons décidé de proposer des modifications importantes au texte. Nous avons voulu distinguer strictement entre les squatteurs et les locataires en difficulté et écarter ainsi tout amalgame. Nous pensons également qu'il est contraire à l'intérêt des propriétaires, comme des locataires d'affaiblir les possibilités d'un accord amiable et d'un règlement de la dette locative sous l'égide du juge qui doit pouvoir vérifier le montant de la dette, la décence du logement et établir un échéancier et des délais de paiement sur la base d'un diagnostic social et financier. Nous pensons enfin que la véritable responsabilisation des locataires résultera d'un accompagnement et d'une prévention précoce des impayés et des expulsions c'est pour ce que c'est, pourquoi j'ai voulu introduire un nouveau chapitre dans la proposition de loi en m'appuyant sur les acteurs du secteur. J'ai proposé d'avancer à deux mois d'impayés, le seuil de saisine des CAPEX de doubler le temps disponible pour la réalisation d'un diagnostic social et financier mais aussi de débloquer de nombreux points techniques pour donner aux CAPEX. Plus de moyens d'agir ainsi, tout en renforçant le volet contre le squat et en luttant contre l'usage dilatoires des procédures par les locataires de mauvaise foi avec André Reichardt. Nous avons voulu donner un équilibre significativement différent au texte et être fidèle à nos principes en termes de respect de la propriété privée des fruits du travail mais aussi de justice et d'humanité. Alors, nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Monsieur Guy Bénard Rochat. Et les membres du groupe écologiste solidarité et territoires ont déposé une motion. Ont distribué sous le numéro 1 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte, en discussion. La parole est donc à monsieur Guy Bénard Roche pour la motion et pour 10 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente. Monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, messieurs les Ministres, chers collègues. Certaines lois marquent une époque du sceau de la grandeur ou de l'abandon. C'est une phrase de Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Dans sa dernière tribune pour nous alerter sur les conséquences de la loi qui nous est présenté la vendant cher collègue, c'est celui de la solidarité. Ce texte se trompe de cible, juge-t-il, comme Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, dans un courrier adressé il y a quelques jours à Gérard Larché, le président du Sénat. Ce sont les causes du mal logement qu'il faut combattre pas ceux qui en sont victimes. C'est une arme atomique qui va donc pas résoudre le problème visé. Mais créer des dégâts collatéraux dans toute la société française subira les conséquences. un bandeau de la solidarité camoufler de manière plus ou moins. Mais définitivement avec une grande violence. Derrière l'érection du droit de propriété comme une valeur absolue. fait d'éviter tout raccourci dans lequel. Certains souhaitent parfois nous enfermer. Je vais le dire d'emblée et sans ambages. Nous ne remettons pas en cause le droit de propriété et sa portée constitutionnelle. La propriété locative doit être et et protégé. D'autant que, comme nous le voyons dans nos communes populaires, on peut être propriétaire et fragilisé par l'âge par la santé par le niveau de revenus. Et dans nos rangs, nous savons aussi que les principes constitutionnels doivent se concilier se concilier de manière équilibrée équilibré. À l'inverse de ce texte qui telle qu'il a été voté par l'Assemblée nationale ne le recherche pas d'ailleurs l'équilibre. C'est donc à nous, ici dans cet hémicycle de faire le travail qui a été commencé par les rapporteurs. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 janvier 1995 a érigé au rang d'objectif de valeur constitutionnelle la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent. Le présent texte quoi que modifié par notre commission pour éviter les amalgames inique entre protection de la propriété des domiciles est un danger. Une fausse solution inefficace et anti-sociale. Il revient à une criminalisation insupportable de la précarité et de la pauvreté. Étudiant d'abord le du droit de propriété sans limite. Je ne ferai face à personne. Si je rappelle combien dans cet hémicycle celles et ceux-ci attachés un droit de propriété absolue en par contre estimé dans un passé récent que l'absolu le était finalement pas tant que ça. Lors de l'étude du texte sur l'ex-patron l'expropriation des biens manifestement à l'abandon. Nous avons bien noté que le droit de ne rien faire de bien resterait sacro-saint quand il s'agit de bien construit fini et entretenu qui pourrait participer à l'hébergement des mal logés mais ne saurait être toléré. Quand une collectivité peut y avoir une opportunité de développement. C'est donc un droit absolu à géométrie variable. La volonté de mélanger domicile local d'habitation locaux ayant d'autres destinations nous pousse sur une pente dangereuse cela déborde l'ambition d'un texte qui n'a que faire de l'équilibre entre les propriétaires, les bailleurs et les locataires équilibre mis en place en 1989. Constamment amélioré depuis et protégé par tous les acteurs institutionnels et professionnels du secteur mais qui sera mis à mal et détruit par ce texte. Une autre hypocrisie la tentative très maladroite et fragile, constitutionnellement d'après l'aveu même du garde des Sceaux de confort, de protection de la propriété du domicile le domicile et la propriété sans protéger de va dire différencier et pour tous les cas affreusement triste et scandaleux de propriétaires de pouvoir intégrer leur domicile, ce n'est pas le manque de protection dans notre droit qui est en jeu mais une méconnaissance des mécanismes de protection. Le président du Haut comité pour le droit au logement, le rappelle dans un courrier adressé aux membres du Sénat. Il semble que la plupart du temps les propriétaires en particulier les plus modestes souffrent plutôt d'un manque de moyens de la justice et d'accès au dispositif de prévention des expulsions. Plutôt que d'un droit inefficace. Venant à cette criminalisation des locataires en difficulté elle est non seulement totalement et des sortes mais inutilement. Car elle ne peut pas apporter une solution à ce problème. Faire porter la responsabilité d'un point de vue pédale aux personnes en difficulté. Que l'État n'a pas pu. Traiter et d'un cynisme rare les mesures d'aides sociales relatives à l'hébergement des familles en graves difficultés économiques ou de logement relève de la responsabilité de l'État qui est parfois trop défaillant. Les collectivités de peuvent se substituer à la puissance publique nationale. Une décision récente du Conseil d'État a rappelé que la carence avérée prolongé de l'État est caractérisé, chambre des territoires. Nous savons combien les collectivités tentent de pallier quelques fois aux manquements de l'État Dobre particulièrement dans les besoins de mise à l'abri quand elles le peuvent, et que l'État les laisse faire. Mais où est ce gouvernement. Où est la politique du logement ben fois danser toujours reporter enlevé du projet séparatisme. C'est l'Arlésienne du président Macron en 2018, celui-ci avait déclaré, je veux que nous puissions apporter à toi à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abris. En 2022, le ministre délégué chargé du logement Olivier Klein a réduit cet objectif au seul enfant et depuis, Monsieur le Ministre. Le locataire reste parce que l'État est incapable de respecter ses propres obligations en matière de droit au logement ou à l'hébergement, c'est une phrase de Claire Hédon, la défenseure des droits qui s'inquiète des conséquences d'une adoption de la loi pour des milliers des personnes déjà sur le fil. J'ai entendu et apprécier les discussions en commission chers collègues qui aura appuyé le besoin de prise en charge des locataires en difficulté via l'établissement d'un bilan social des locataires, mais qui pourra effectuer ces bilans ou sans les moyens pour les préfectures d'accompagner ces personnes en difficulté. Les débats de la haine ont permis de rappeler le manque de moyens pour les travailleurs sociaux du 115 le manque de places d'hébergement d'urgence chaque soir en France 5000 personnes appellent envers le 115 dans l'espoir d'une place en hôtel ou en foyer d'urgence à Marseille où 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté. À peine un appel sur 3 aboutit. Où est l'État et puis toutes ces histoires aussi tristes les unes que les autres de petits propriétaires qui sont dans l'impossibilité de récupérer leurs domiciles occupés illégalement, sans souvent le reflet de méconnaissance ou d'action des services de l'État médiatique et insupportable. Toutes ces situations ont été résolus, sans nécessité de modifier la loi. Étant. Capacité. Étant capable de trouver un chemin pour protéger à la fois les propriétaires les locataires les personnes mal logées ou à la rue. Les moyens de protéger les petits propriétaires existe des mesures de protection équilibré pour les propriétaires et les locataires pourraient être à forcer comme la garantie loyer. Mais rien dans l'écriture du taxe ni même sa réécriture moi délirante par la commission de notre assemblée ne montre que le but de cette loi et la protection de ces petits bailleurs parfois démuni face aux démarches. Le but affiché punitif. La conséquence la punition de familles en difficulté une criminalisation de ceux qui subissent la précarité, ceux qui souffrent du mal logement et pour qui, peu de solutions ça offertes, plus de 4.000.102 personnes sont mal logées. 300.000 sont sans abri dans 42.000 enfants les chiffres sont édifiants. Les causes sont multiples, complexes, mais la crise actuelle inédite entraîne une accélération de la paupérisation des policiers populations fragiles. Les solutions à cette détresse qui poussent les personnes dans la rue, dans les situations de payer ce que Proposition de loi appelle des occupations frauduleuses sont absents du texte de loi. La notion de pénalisation de prison pour des problèmes d'impayés est une notion insupportable Vous De plus, vous ne pouvait plus payer votre loyer, votre bail résilié et pourtant vous occupez encore votre logement faute d'autre solution que la rue en prison la prison pour dettes est de retour dans notre République. Serions-nous prêts à ériger cette dette comme la plus criminelle au sein de notre société, au-delà de, de la réflexion insensé. Ils vont l'insolvabilité de loyer comme différente des autres elle solvabilité. Quelle est la finalité de cette pénalisation par une peine d'emprisonnement toute sanction financière sous forme d'amendes aura aussi pour conséquence de créer un cercle vicieux maintenant les occupations, dans une précarité à part une valeur symbolique depuis édition qui sera gagnant que gagnera le propriétaire qui sera qui aura encore moins de chance de recouvrer sa dette. Le président du Haut comité pour le droit au logement, nous la rappelé. En privilégiant l'expulsion les propriétaires auront beaucoup moins de possibilités de recouvrer leurs dettes et locataires rejoindront les rangs des sans-domicile-fixe ou des sans-, abri, la précarité et le problème de base, avec un contexte actuel incertain. L'inflation, l'accroissement des contrats précaires. L'augmentation des factures énergétiques, la diminution des ah d'habiter de chômage. Les situations de défaut de paiement se multiplieront les dispositifs de mise à l'abri d'hébergement d'urgence d'application du Dalo ne sort pas suffisamment mis mis en oeuvre et sort pourtant les solutions que vrai texte sur le sujet aurait dû prendre en coque tout au contraire des dispositions de ce texte dans la Fondation Abbé Pierre estime qu'elles vont provoquer jusqu'à 30.000 décisions d'expulsions supplémentaires soit autant de personnes qui risquent de se retrouver à la rue. Mes chers collègues. C'est avec une certaine fascination que j'observe la tentation, disons-le, un peu démagogique de positionnement sur le droit de propriété que personne, encore une fois ne remettent en cause ses positionnements fortement affirmé et défendu par certains ici sont pourtant variable, comme j'ai déjà pu l'évoquer dans le cas de l'expropriation des biens hors d'état d'abandon manifeste un jour ce droit de propriété est absolue dont il ne l'est pas. C'est notre devoir de garantir les droits et la protection des plus vulnérables. Si la loi telle qu'elle nous est arrivé de l'Assemblée est caricature dans la surenchère, de déséquilibre de pénalisation à outrance faisant un amalgame pour le coup coupable entre protection de la propriété protection du domicile autre squat et incapacité de payer si je remercie les rapporteurs.

Madame pro-caisse si. Ah vous n'êtes pas rapporteur donc c'est bon. Même Catherine Procaccia contre la motion pour 10 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Ce soir, c'est un anniversaire. Hé oui. Je ne peut que penser à la nuit du 31 janvier 2007. Il y a quasiment 16 ans jour pour jour, j'étais bien seul dans cet hémicycle pour parler des squatters. Des sites internet qui déjà à l'époque délivrer un mode d'emploi. Et j'expliquais à mes collègues. De différents bancs qu'il fallait aussi penser à la personne, locataires ou propriétaires qui se retrouver à la rue grâce à squatter. Dans la nuit, j'ai reçu des manifestants. Des manifestants du DAL, le droit au logement de jeudi noir. Et ils ont convenu avec moi que mon amendement qui est devenu l'article 38 de la loi Dalo était acceptable. S'il se limitait au squat de l'habitation principale, telle est l'histoire de d'un amendement 38. Hélas, cet amendement que vous avez de nombreuses fois évoquées, monsieur le garde des Sceaux a rarement été mises en oeuvre et il a été pendant très longtemps très peu appliquée par les préfets. 11 ans après. Autre petits pas quand, soutenu par le rapporteur de la loi Elan le Sénat puis la CMP ont adopté mon amendement qui précisait que la trêve hivernale ne s'appliquait pas aux squatters là contre l'avis du garde des sceaux de l'époque qui disait que ça tombait sous le sens mais une fois que ça a été écrit, c'est aller beaucoup mieux. Comme j'ai pu le dire en 2021 à Dominique Estrosi Sassone et Henri Leroy, quel bonheur de voir la relève enfin assuré que je n'étais plus là seule a souligné les inéquités du droit pour cet acte d'ailleurs si le texte de 2021 comme l'a dit notre rapporteur. Avait été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, nous n'aurions pas aujourd'hui besoin de ce nouveau débat. Il ne faut pas oublier non plus que la notion de squat a été étendue aux résidences secondaires depuis la loi ASAP et que depuis un an, l'intervention des commissaires de justice devrait faciliter la procédure. Et quel plaisir monsieur le garde des Sceaux de vous entendre reconnaître que le squat est un délit. Nous n'avons pas toujours eu le plaisir en tout cas au Sénat d'entente des gardes des Sceaux l'affirmer. À mes collègues écologistes qui remettent en cause cette PPL j'affirme que amender avec beaucoup de circonscriptions circonspection des formations. Par nos deux rapporteurs elle établit bien la distinction entre squatteurs et locataire et je leur demande, avez-vous été un jour réellement en face d'une personne qui, à son retour de l'hôpital. Ou d'un voyage ne peut plus rentrer chez elle et à laquelle on demande de justifier que c'est bien son domicile alors que là. Non demande rien squatters et qui est là tous ces documents peut être détruit à l'intérieur de son domicile. Je remercie à cette occasion la commission qui a repris un de mes amendements. Qui avait d'ailleurs été adoptée en 2021 par le Sénat qui prévoit que le préfet peut solliciter et doivent solliciter l'administration fiscale pour les titres de propriété ou d'occupation légale logement puisque ce ne sont pas que des propriétaires, mais aussi des locataires qui parfois ne peuvent pas rentrer chez eux. Mes collègues porteurs de la motion d'irrecevabilité, argue que l'on ne peut qu'on ne pénètre pas dans le domicile d'autrui par plaisir et que chacun doit disposer d'un domicile descend. C'est un argument que nous sommes nombreux à comprendre mais je demande, est-il normal dans ce cas que les cellules les serrures soit. Tout comme très rapidement le nom de la du titulaire de la quittance d'électricité et que les squatteurs refuse de partir quand les propriétaires ou les locataires légitimes leur demande et même après un jugement de justice quand il ne dégrade pas les lieux. Est-il normal que les décisions de justice rendues à la faveur des propriétaires du logement parfois après plusieurs années ne soit pas appliquée. Ce laxisme ne fait qu'entretenir les squatteurs dans leur sentiment d'impunité. Et non Monsieur Bénard Roche tous les cas ne sont pas réglés. Des cas que nous voyons à la télévision ou dans la radio ne sont pas tous les cas et ils ne sont pas si exceptionnel que ça. Le droit au logement existe, je l'affirme mais il doit s'appliquer à tous y compris aux titulaires du logement c'est mon intime conviction. J'estime aussi que les propriétaires évincés par les squatteurs devraient aussi pouvoir être relogés est réellement indemnisés. Si le préfet décide de ne pas exécuter une décision de justice. Voter la motion d'irrecevabilité de mes collègues ce serait rayé les avancées attendues depuis longtemps comme l'accélération de la procédure contentieuse locatives ou celles apportées par la commission qui distingue bien Water bien Water locataire qui ne plaît plus et volontairement qui ne perd plus et qui libèrent les propriétaires de leurs responsabilités pour l'entretien de biens auxquels ils ne peuvent plus accéder. Et s'il y a je nous le savons tous, des propriétaires indélicats. Il y a aussi des locataires indélicats rééquilibrer les droits permettra, je l'espère, de remettre sur le marché de la location de nombreux logements toutes ces raisons font que le groupe républicain que je remercie de m'avoir donné la parole pour défendre ce texte votera contre la motion les recevabilité. Mes chers collègues, nos collègues souhaitent opposer l'exception d'irrecevabilité, considérant que la proposition de loi contrevient nos grands principes et notamment à l'objectif à valeur constitutionnelle, l'accès au logement. La commission ne partage pas cette analyse. Le texte issu de ces travaux contient plusieurs dispositions qui viennent justement prévenir les expulsions et améliorer l'accompagnement social. Les locataires en difficulté donc la commission a émis un avis défavorable. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, je le ministre. Merci madame la présidente. Ce soir, après la séance j'irai m'installer chez Monsieur Avec toute mon équipe. Et immédiatement je franc sorte de changer les serrures. Et comme le font certains squatters je mettrai une petite affichette à la fenêtre. Pour vous dire que si jamais, par effraction. Vous voulez récupérer votre bien. Je vous ferais poursuivre on marche sur la tête. On marche, on marche sur la tête. Il y a il y a des jours qui ont bossé toute leur vie je prenais tout à l'heure l'exemple de cette femme qui part à l'Epad. Et alors vous savez il y a des professionnels de d'abord il y a sur Internet comment squatter un on a vu il y a tout un tout un truc qui s'est mis en place mais on met un petit morceau de papier sur la porte et quand on constate qu'il a pas bougé. Ça veut dire que c'est inoccupé parce que la dame est as pattes parce que le, le couple est parti en vacances et puis d'autres viennent là où. Oui c'est une infraction et ça doit être une infraction. Je vous ai fait plaisir madame la sénatrice, c'est franchement ce que je pense. Je sais pas ce qui a pu être dit par certains de mes prédécesseurs Maeva vous rentrez chez les gens, ça devient votre domicile, vous n'avez plus le respect de rien. Moi je veux bien. Hé oh non

Vous aurez votre temps de parole. Merci. Alors. Je vais consulter le Sénat sur l'exception d'irrecevabilité. Monsieur Savoldelli. Merci madame la présidente. On va passer un moment avec. Les convictions les passions des uns et des autres. Mais monsieur le garde des Sceaux. Moi je vous demande pas de venir chez moi.

Mais bon on voit votre récit de venir chez un parlementaire enfin franchement. Le sujet est trop important. Donc je vais vous donner d'explication. Il y a évidemment une argumentation opposable à ce que je veux dire. Mais j'ai pas partir d'un récit d'un roman de je ne sais quelle histoire. Voilà, je vous dis mais cette opposable. Moi je pense que la question des recevabilité, nous allons la voter je vous dire pourquoi et qu'on va y revenir après avec la question préalable de manière calme et extrêmement respectueuse. Il y a un problème de déséquilibre, à mes yeux, aux yeux de notre groupe. Peut-être que nous avons tort entre 2 droits qui sont à la fois. Les droits attends Et les droits fondamentaux garantis par la Constitution, dans lequel il y a le droit au logement. Nous pensons nous pensons et ce que de de nous de penser. Que il y a un déséquilibre dans la façon dont est abordée la question des squats et des impayés avec un mélange de genres, qui n'a pas lieu d'être et un déséquilibre sur la question des libertés et des droits fondamentaux entre le propriétaire et le locataire, c'est un point de vue quand même qu'il s'entend et c'est pourquoi notre groupe soutiendra recevabilité qui est proposé par notre collègue nos collègues du groupe au cours pour Europe Écologie Les Verts. Voilà et tranquillement. Merci madame Artigalas. et c'est à juste titre que cette motion rappelle dans son objet. La décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 1995 et le vent aura d'Oran d'objectif de valeur constitutionnelle la possibilité tout pour toute personne de disposer d'un logement décent. Ceux qui prendront la peine de relire cette décision verront que les sages cite des passagers du préambule de la Constitution de 1946 qu'il paraît essentiel de répéter ici ce soir la Nation assure à l'individu à la famille les conditions nécessaires à leur de développement et elle garantit à tous le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence y compris lorsqu'une personne un être humain se trouve dans l'incapacité de travailler en raison de son état physique ou de la situation économique. groupe s'interroge sur un point particulier, l'Irak, les rédacteurs de cette proposition de loi, estime-t-il que le fait de prévoir une peine d'emprisonnement pour punir quelqu'un de marrant encore dans son logement après avoir dû faire face à l'impossibilité d'en payer son loyer et la manière la plus adéquate pour notre dation d'assurer à l'invite individus à la famille et les conditions nécessaires à leur développement des moyens convenables d'existence. Parce que nous trouvons cette proposition de loi ni recevable ni acceptable et encore moins soutenable pour toutes les Françaises et tous les Français, notre groupe votera cette motion et parce que aussi cette proche ce projet de loi est déséquilibré introduit un déséquilibre.

d'une primauté soi-disant absolue du droit du, du droit de propriété et invoqué le logement décent comme si c'était un permis de et un sauf conduit à bafouer les droits les plus élémentaires du, du droit de propriété, c'est quand même une drôle d'interprétation parce que monsieur. Vous manquez pas de de de référence. C'est quand même le 1er des droits qui a été affirmé à 1789 c'est pas rien, c'est pas rien, au même titre que la sûreté mes petite que l'égalité de l'homme en droit au même titre que la liberté, la récente ça l'oppression. Alors maintenant vous vous y invoqué le droit au logement qui certes est tout à fait. Admissible mais il y a quand même une primauté du droit, du droit dans son exercice du droit au logement que vous veniez absolument et invoqué la crise du logement à tout propos, qui est une réalité

et qui a figure en rédaction et qui a figuré à l'article 17 de des créations, droits de l'homme c'est quand même quelques rappels qui sont nécessaires à ce stade de la discussion. Merci cher collègue alors je. Oui, Monsieur le Ministre, pardon. Je voudrais je avais oublié. Je suis vraiment désolé. Non je voulais madame la présidente. Je veux rassurer tout le monde répondre très brièvement à votre interpellation. Monsieur le sénateur, en réalité. J'ai pas voulu vous offenser mais ce que j'ai dit sur un ton un peu bada peut être. N'aurais-je pas dû. Mais c'est exactement ce qui se passe. Le le le droit au logement. Dont vous faites et le fervent défenseur il existe mais c'est pas, pousse-toi là que je m'y mette.

Vous l'avez pris pour quelque chose. D'offensant et si c'est le cas je je vous présente mes excuses mais, mais c'est ça le squat, c'est je je je trouve un logement vide, il n'est pas à moi au nom du droit au logement, je je vais au fond mis installer j'interdis ensuite aux propriétaires de récupérer son bien. Bon je sais pas la propriété c'est pas sale. C'est pas moche c'est consacrée aussi par notre Constitution. Il faut le rappeler et moi je trouve que ce texte il a le mérite d'être un texte équilibré. Voilà. Entre naturellement le droit au logement mais également le droit constitutionnel à la propriété privée et les situations que nous avons vu ces temps derniers, au travers d'un certain nombre de reportages sont à proprement parler. Inacceptable. Inacceptable, vous avez ces jours derniers, des gens qu'on a vu qu'ils dorment sur leur terrain dans leur caravane. Parce que la part qui est le leur. Ils ont bossé toute leur vie est occupé par des gens qui ont décidé que le droit au logement surpassé tous les autres droits enfin pardon, mais moi je ne peux pas être sur cette position là. Merci. Alors je vais consulter le Sénat sur l'excès. Dure 10 recevabilité. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte, en discussion l'avis de la commission et l'avis du gouvernement et contre la motion. Donc il est pour la motion. Qui est contre. Qui s'abstient. La motion n'est pas adopté. Nous passons la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Madame Éliane Assassi. Les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Ont distribué sous le numéro 6 tendant à opposer la question préalable au texte, en discussion et la parole est à monsieur Pascal Savoldelli pour la motion et pour 10 minutes.

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues. Je commence bien. J'ai peur parler le président de la République. 2017. Emmanuel Macron, il déclare.

Dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité. C'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi, fin de citation. Une question donc. Quelle est la place qu'il accorde. Cette proposition de loi à la dignité des plus vulnérables. Depuis la création du droit au logement inscrite dans la Constitution qui permet l'expulsion sans jugement du domicile occupées illicitement. Les réformes successives en matière d'expulsions sans jugement du domicile occupées illicitement se sont renforcées. D'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure. Ces réformes ont été alimentées de faits divers. Pour beaucoup, je m'excuse beaucoup sur médiatisée de l'an, l'impression que les phénomènes du squat et et des impayés de loyers d'ailleurs injustement assimilés depuis tout à l'heure injustement allez on fait un amalgame entre les squats et les impayés de loyers aurait pris une ampleur considérable. On serait face à un tsunami. On serait dans un quasiment dans un régime d'occupation avait ce qu'elle dit. Et pourtant, mes chers collègues. Nous sommes loin d'être laxiste en la matière. Mais ces phénomènes je mais ce qui reste quand même très rare. Certains ne veulent pas le reconnaître le squat. Et pas toujours Et pas toujours est loin d'être la première issue voulue par les personnes. C'est une solution forcé. Qui découle de l'incapacité de l'État. Alors là, bon moi je veux bien qu'il faille pas en parler. Mais à la mise à l'abri à l'accès au logement de tous. Vous me direz, monsieur Misca si je je je je me trompe, je crois que sur l'exercice 2022, vous avez construit 84.000 logements sociaux, c'est ça. Il dit oui donc c'est vous dire que, on dit la même chose. Par contre, 84.000 logements sociaux. Quand on regarde, il faudra à peu près en construire 150.000 pendant 10 ans tous les ans. Vous venez d'envoyer une missive aux préfets, sur la question du froid avec les préfets et cetera. Je vais vous parler tout à l'heure de combien de temps on met à avoir un hébergement d'urgence, 75. Mais vous le savez donc. Donc pourquoi je vous dis tout ça parce qu'on ne peut pas ignorer cette question des réponses de l'État. Si on veut pas de gens à la rue et privé du droit et il convient de souligner juridiquement que l'occupation illicite d'un bien immobilier portent le plus souvent une atteinte réparable droit de propriété. Le propriétaire peut déjà obtenir une indemnisation satisfaisante des loyers impayés ou des dégâts causés par les occupants sans droit ni titre, pourquoi cette loi fait l'impasse sur des dispositifs déjà existants. En fin de compte l'enjeu de cette proposition de loi et d'élever le droit de propriété à finalité lucrative au rang de valeur suprême. Voilà la question, et c'est normal qu'on en débatte. Une valeur qui, aux yeux de ce texte doit primer sur tous les autres principes y compris celui de la sauvegarde de la dignité humaine car oui. Le but avoué de cette proposition de loi et d'aggraver le déséquilibre de la relation entre le bailleur et le locataire et au détriment de ce dernier et a tendance, le mot est dur, le mot est dur mais on y viendra à criminaliser les locataires les plus en difficulté face aux intentions de cette proposition de loi qui ne sont pas ou peu en adéquation avec les réalités économiques et sociales de notre pays. Je pense qu'une piqûre de rappel s'impose, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste dénonce d'ailleurs l'incapacité de l'État à respecter ses obligations en matière de droit au logement. Aujourd'hui, je vous le dis. L'urgence est d'éviter que davantage de personnes et de familles en situation de précarité se retrouvent à la rue. Nous voulions pas qu'en France ce n'est qu'une fois tous les cinq jours qu'on peut être logées par le 115 c'est ça. Monsieur le Ministre. Non, c'est beaucoup moins. Je vais vérifier dans mon beau département, le Val-de-Marne, si c'est moins OK. Le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste est convaincu que prévenir les drames humains. Tout en protégeant le droit des propriétaires. Donc, n'opposons pas les choses, regardons ce qu'on appelle l'intérêt général. Nous pensons nous qu'il faut remettre sur pied la garantie universelle de loyer. Voilà, de renforcer les moyens d'hébergement et de relancer la construction de logements sociaux. Voilà tout l'inverse de ce qui est proposé dans cette loi, mes chers collègues, nous devons nous rendent compte de la gravité de cette proposition. si on la vote on va appliquer pour la première fois des locataires en situation d'impayés de loyers. Des dispositions habituellement réservé aux occupation illicite résultant d'une intrusion avec à la clé. Avec à la clé une peine de prison. Ah bah c'est marqué vous le dites. Et moi je vais vous dire nos prisons. J'espère que vous êtes d'accord avec moi monsieur le garde des Sceaux sont plus que surpeuplée. J'apprends par exemple que dans la plupart des prisons on atteint des taux de surpeuplement anneau de 140 à 160%. C'est pas faux non plus, ça fait quand même pas mal de vérité quand même avec qui sont quand même ici exprimer et sous le prétexte tournées de protéger les petits propriétaires face au squat de leur domicile pourtant déjà puni par la loi d'un an de prison et de 30.000 euros d'amende et d'une expulsion sans jugement en 48 heures. La proposition de loi s'attaque en réalité à toute personne, toute personne en situation de Provoté où le mal logement ou confronté à un accident de la vie en plus d'être un cohérente avec les intentions affichées. Le gouvernement en matière d'expulsions de logement et de lutte contre les marchands de sommeil, tout ça, ça passe à la trappe. On en parle pas et aujourd'hui et ça a été dit par la fondation de l'abbé Pierre, il faut construire 150.000 logements, donc l'absence de la politique gouvernementale et aussi au coeur du débat que nous avons aussi ce soir mais aussi. Pas excusez-moi d'en parler. Ce c'est pas ça va peut-être être une sorte de cavalier législatif, mais dans la question du logement, il y a la question de l'autonomie financière donc il y a la question des salaires. Ouais bah ouais elle s'invite aussi dans cette discussion-là. Et ouais c'est vrai du point d'indice dans la fonction publique, et caetera. Il y a l'inflation, c'est vrai que non mais d'accord monsieur Dupond-Moretti. Mais vous, vous pouvez aller chez l'habitant. Je vous invite à la maison, mais vous avez pas de problèmes financiers quand même pour avoir un logement, on est bien d'accord OK Donc il est indiscutable que les retards de loyers si il n'y a pas des efforts dans ce domaine, il va y avoir mes chers collègues. Plus de plus en plus de retards de paiement des loyers qui vont exploser.

Il va y avoir un problème d'impayé très rapidement d'ailleurs Monsieur le Ministre du logement. Je vous le dis par exemple une proposition constructive, aurait été ici de relever l'APL décharge là on va aider les gens les plus modestes à pouvoir subvenir au paiement de leur loyer. Vous savez le poids que prennent les charges dans la question du coup pour payer son loyer, donc voilà je voulais vous dire que on est aussi dans une situation où on assiste à un nombre de coupures. Ou de baisse d'énergie en terme de coût pour l'eau pour l'énergie. Franchement c'est pas le moment de de de mètres cette loi là au moment où il y a tant de gens qui vont être exclus par nature puisque de toute façon ils vont avoir des factures qui ne peuvent pas payer. être, on va se retrouver dans une situation excusez-moi, je considère comme assez explosive. Et n'oublions pas que la privation domicile peut être également. Alors je sais que là on, on va me dire ça fait un peu de sociologie des sciences humaines mais bon. vous êtes cavalier comme ministre hein franchement. Allons-y, qui me dit. Allez vas-y parle de ça, bah je vais vous en parler. Ouais. Le fait de pas avoir de domicile sur le garde des Sceaux. Ça peut être une étape de désaffiliation sociale. Vous le savez bien et qui conduit aux formes les plus graves d'exclusion. Et mes chers collègues. Comme le souligne la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt en date du 17 octobre l'arrêt dit Winterstein France la perte d'un domicile entraîne souvent des atteintes à d'autres droits cruciaux je cite pour l'identité de la personne l'autodétermination de celle-ci son intégrité physique et morale, le maintien de ces relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position au sein de la société, donc on est sur un sujet extrêmement important. Ainsi la procédure pénale visant à réprimer le comportement des occupants en cas de violation de domicile ou dégradations de biens peut entraîner des interpellations. Mais elle ne peut en aucun cas, constituer un mode d'expulsion. Pourtant, l'article premier hein. Ah de la proposition de loi en permettant que le délit de violation du domicile soit constituée. Lorsqu'une personne pénètre légalement dans un logement mais il maintient illicitement autorise un recours plus large et sur une durée presque illimité de la procédure de flagrance une procédure pénale qui est ici un mode d'expulsion. Et encore une fois nous sommes face à une disposition ni nécessaire ni proportionné, notre groupe dénonce ainsi une proposition définitivement dangereuse et ceux du et sur de multiples droits fondamentaux et en effet, comme le rappelle le président de la convention nationale de la Ligue des droits de l'homme. Monsieur Burguburu. Cette proposition de loi fait peser sur les associations qui travaillent auprès des personnes mal logées ou sans abri, le. Délit de propagande ou de publicité visant à inciter à l'occupation sans titre. Nous craignons pour leur liberté d'expression.

madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, L'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est clair. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression. Même si le droit de propriété a une valeur constitutionnelle. Nous sommes toujours face à des violations de domicile et d'occupation des biens immobiliers par des squatters. Pourquoi vouloir revenir sur ces acquis de la révolution, c'est paradoxal. Et une fois encore, alors que nous tenons. À obtenir plus de justice parce que lutter contre la spoliation de la propriété, c'est obtenir plus de justice et de fermeté. Vous nous opposer de l'humanité, comme si les deux étaient incompatible alors que c'est l'inverse, comme si nous devions faire preuve d'humanité envers ceux qui ne respectent pas la loi au détriment du droit des propriétaires. Oui l'humanité quand on spolie les personnes. En effet, de quel propriétaire Palm on nous et nous en avons parlé, vous en avez parlé. Monsieur le ministre et j'étais ébahi de voir que pour une fois, nous étions d'accord. Nous parlons de retraités qui ont économisé toute leur vie. Nous parlons de jeu de propriétaires qui se sont endettés pour s'offrir un trois pour y fonder une famille nous parlons de famille aussi, à qui on vole leur souvenir, nous parlons de rêves brisés par des individus qui ne pensent qu'ils se pensent parfois au-dessus des lois. Le droit au logement, ce n'est pas celui de voler ou de détruire. C'est tout à fait la verse, nous parlons de ces familles qui souvent. Utilisent les failles du droit et je veux remercier souvent la presse qui se fait l'écho de de situations dramatiques qui ont été évoqués ici. Dans places à certains. Nous parlons souvent propriétaires bien modeste. Je voudrais vous citer quelques exemples en 2020 après un tour du monde écourtée pour des raisons de santé. Maryse et Pierre avait voulu retourner vivre dans leur maison louée le temps du voyage mais la nouvelle habitante refusé de quitter les lieux. Elle a ensuite cessé de payer le loyer. Les chars il y a quelques jours à Pamiers dans l'Ariège. À 75 ans, Georgette pensé vivre une retraite heureuse dans une petite maison qu'elle s'est haché il y a plus de 20 ans en centre-ville. Et elle explique. Aujourd'hui dans la presse que l'homme qui avait mené les travaux de rénovation refusé de quitter les lieux à Mazingarbe dans le Pas-de-Calais, une maison d'un riverain squattée saccagée pendant plusieurs jours juste après les fêtes de Noël. Pire encore, les propriétaires étaient même séquestré. Les squatters sont même revenus à 2 reprises ensuite pour voler de la nourriture dans le réfrigérateur de la victime. Ça peut peut-être vous faire sourire, mais ces situations humainement dramatiques Mégane qui avait hérité d'une maison squattée. Après s'invite dans la Somme, en octobre 2022, elle avait ému les Français en parlant de son combat pour la récupérer, s'installer, d'installer une tente d'accrocher des banderoles et des pancartes devant sa maison pour dénoncer l'absurdité de la situation une propriétaire de 24 ans à la rue et le squatteur à l'abri. Elle espérait faire évoluer la situation avant la fin de la trêve hivernale, le premier avril 2023. Elle dénoncé la lenteur administrative concernant le jugement d'expulsion et en ce début d'année son constat est amer, je la cite pour la maison. Malheureusement, il n'y a aucun changement, puisqu'il n'est pas expulsable avant la fin de la trêve hivernale, évoque-t-elle. Oui l'humanité. Malheureusement ces cas médiatisés ne sont pas les seuls, il y en a de nombreux autres et militer pour un logement digne. Et compréhensible, excusez la la destruction ou la spoliation du bien d'autrui pour moi ne l'est pas et ce je trouve ça à la fois incongru et injuste. Ces atteinte manifeste au droit propriétés sont inacceptables. Alors que la France n'est malheureusement pas un cas isolé puisque malheureusement des voisins européens connaissent des parcours. Similaires aux nôtres. Mais les propriétaires victimes de ces occupations illicites qui font pourtant valoir leur bon droit se trouvent dans des situations d'impuissance à laquelle il est de notre devoir de répondre et les mères aussi sont démunis face à ces situations. Au choc s'ajoutent les frais de justice les réparations et les délais d'inacceptable eu égard aux différentes situations dans nos circonscriptions concernant ces occupations illicites. Il est logique que nous, représentants du peuple français représentant des communes, nous fassions ce qui est en notre pouvoir pour mieux protéger nos concitoyens. Nous ne sommes pas seulement face à des faits divers. Nous sommes face à de véritables drames. Nous sommes surtout face à une réalité. Le droit n'est pas respecté, les propriétaires se sentent souvent démunis, voire abandonnés par les pouvoirs publics. Pire, ils estiment que le droit n'est pas de leur côté et qu'à l'inverse il protège ceux qui occupent une maison en toute illégalité. Ces situations d'anormal et inadmissible défient ouvertement l'autorité de l'État et sa capacité à garantir l'ordre public. Ce n'est pas acceptable dans notre État de droit. Si l'État ne remplit pas ses obligations les plus élémentaires, comme celle de faire cesser les atteintes aux droits de propriété. Alors notre contrat social est en péril. Et c'est pourquoi il est de notre devoir de parlementaires d'agir. Je ne peux que regretter que le gouvernement perdre autant de temps sur cette question si grave parce que nous nous sommes retrouvés en 2020 face à ce débat et vous avez rejeté. Les propositions que nous avions pu faire. Et voilà des années qu'avec ma famille politique, les républicains nous formulons des propositions qui sont systématiquement rejetés rangé dans les archives ou même à ce moment-là reprise mais tardivement par la majorité présidentielle et d'ailleurs je voudrais saluer les travaux de notre collègue, ancien député Julien Aubert et de notre collègue Dominique Estrosi Sassone qui ont travaillé sur cette question et dont les propositions ont été rejetées en 2020. Pour mémoire en 2019, Julien Aubert et moi-même alors parlementaire nous avions déposé une proposition de loi visant à augmenter le quantum des peines portées à 3 ans et des peines de prison jusqu'à 45.000 euros d'amende. Pour ces délits et accroître la capacité des pouvoirs publics à évincer les squatteurs dans des délais rapides mais aussi à qualifié ce délit ces propositions présentées au moment de l'examen de la loi, on va l'appeler la loi Wargon ont presque toutes été retoqué et je le regrette que de temps perdu que d'injustice depuis le 1er décembre dernier, les députés les républicains devaient inscrire un texte sur ce sujet. Malheureusement, la majorité présidentielle comme souvent a souhaité. Reprendre une grande partie de nos travaux et les inscrire sur leurs propres textes au lieu de faire un travail commun avec ce que nous avions proposé. Mais bien sûr. Ce qui compte c'est l'intérêt des Français. Je regrette mes chers collègues, sur ce sujet comme sur d'autres sujets. La majorité présidentielle perdent du temps avec des stratégies politiques et des récupérations politiciennes parce que tout ce temps perdu, ce sont des injustices qui court, ce sont des situations de détresse auprès des Français et tout ça pour revenir avec tant de retard sur ce que nous avions déjà proposé. Je dois dire que nous sommes constants sur ces questions. Et que nous soutenons ce texte avec les modifications apportées par la commission des lois et je veux remercier notre collègue le rapporteur André Reichardt. Et c'est pourquoi je vous invite à vous opposer à cette question préalable. Parce que notre souci c'est de protéger davantage les Français les propriétaires c'est de lutter aussi contre le recours à une justice privée ce qui est la conséquence regrettable d'une action publique souvent impuissante est considéré comme injuste. Comment ne pas être révolté, lorsque nous avons tous vu des reportages. Ou des familles se retrouver devant un bien qui était occupé saccagé dégradé pendant des années avec des frais de justice. Cette situation s'est produite à Marseille dans dans le 12ème arrondissement je, je me souviens très bien d'avoir reçu les, les propriétaires de cette maison et lorsque l'évacuation a enfin eu lieu. Hé bien eux qui avaient été si seul pendant toutes ces années ont vu les services sociaux, venir au secours des personnes qui les avaient spoliés qui leur avait volé tous leurs souvenirs qui avait dégradé la maison de leur enfance et pour lesquels ils n'avaient plus aucun recours. Autant on peut prendre en compte des situations de mal logement. Ce qui est tout à fait normal, mais là je trouve qu'il y a à la fois une injustice et un aveu d'impuissance. Et comme une prime aux personnes qui triche et qui vole parce que c'est du vol et qui spolient ces honnêtes gens. Et c'est la raison pour laquelle je dis que d'ailleurs ce texte que nous examinons aujourd'hui il y a parfois pour certaines personnes, des décennies de souffrance des citoyens honnêtes qui ont été broyées par les travers du droit il y a même une économie parce que il y a des personnes qui viennent voir ces ces ces pauvres Français spoliés et qui leur propose de racheter leur maison à vil prix parce qu'ils ont les moyens parfois peut être avec. Des gros bras ou. De faire de faire pression sur les squatteurs pour qu'il parte et ils rachètent ses bien à vil prix, tout ça est particulièrement injuste et c'est la raison pour laquelle il faut protéger nos concitoyens et surtout ceux qui respectent le droit toutes ces personnes qui aujourd'hui sont d'un déficit des difficultés nous regarde. Soyons leur porte-parole et surtout, espérons qu'avec une confiance que nous pourrons redonner dans la propriété, hé bien ces personnes retrouveront confiance pour pouvoir mettre leurs biens et le louer pour que la crise du logement justement diminue et qu'elle ne s'aggrave pas par les incertitudes qui pèsent sur les propriétaires et c'est sur des mesures simples que jeu de mot demande mes chers collègues, de vous engager et de vous rappeler que si nous sommes là c'est pour oeuvrer pour que les Français soient mieux protégés pour l'intérêt général

La vie de la commission. Monsieur le rapporteur. Ce sera un avis défavorable. Madame la présidente. Nos collègues du groupe CRCE rappelle à juste titre l'ampleur de cette crise du logement. Ils évoquent. À juste titre le chiffre de 300.000 sans-abri, 3 millions de logements vacants. Ces données démontrent s'il en était besoin, la nécessité de réformer le marché du logement. Mais beaucoup de propriétaires hésitent à mettre leurs biens en location parce qu'ils craignent d'avoir toutes les peines du monde à le récupérer en cas d'impayés de loyers. La proposition de loi vise précisément à rétablir la confiance pour ramener des logements sur le marché de la location et cette PPL vise également à lutter avec plus de fermeté contre le phénomène du squat qui est un phénomène distinct je rajouterai enfin. Ce cher collègue ça vaut chère Pascale il y a 97 amendements à examiner un certain nombre, viennent du groupe CRCE je m'apprête à donner un avait un certain nombre d'avis favorables qui vise précisément à aller dans le sens que vous souhaitez, pourquoi voulez-vous qu'on arrête là la discussion alors. On peut peut-être avancer pour le bien être à la fois des locataires et des propriétaires dans ce pays. Oh moi très franchement un avis défavorable je vous inviterai même à retirer cette demande de questions préalables. Merci. L'avis du gouvernement. Monsieur le Ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Notre avis sera aussi défavorable d'abord parce que on l'a dit, ce texte est équilibré, à aucun moment il mélange. Les squatteurs et les personnes en situation d'impayés de loyers. À aucun moment et. Le texte sera encore amélioré et il a déjà été très largement par le travail préalable de la de la commission, notamment sur la question de la bonne foi vous soyez vous-même de bonne foi, si vous lisez ce texte. Vous savez bien qu'aucun locataire de bonne foi finira en prison pour pour impayés de de loyer, enfin j'ai quand même vous donner quelques réponses sur la situation ce soir c'est 203.000 places d'hébergement d'urgence qui sont ouvertes dans ce pays, c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint par le passé par aucun des gouvernements précédents c'est 5,7 millions d'euros qui est dépensé sacs chaque soir par ce gouvernement pour mettre des personnes à l'abri et et ce chiffre, il est extrêmement important. Il est malheureusement difficile. À apercevoir mais je peux vous assurer que c'est un travail quotidien que nous menons avec toutes les associations pour arriver à cette situation, le plan logement d'abord lancé par le gouvernement précédent, c'est 440.000. Personnes qui ont quitté la rue pour aller dans un logement aucun gouvernement. N'avait fait. Un une action aussi forte pour sortir les gens de la rue et ça fait partie des engagements du gouvernement demain lors du conseil des ministres se fera une communication sur le plan logement d'abord de et, je dirais, comme je le fais tous les ans à la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Oui pour dire que le mal logement est est un mal insupportable, oui le mal-logement est un mal, sur lequel nous travaillons, nous travaillons depuis des années et une dernière chose comme maire ou ex-maire de Clichy-sous-Bois largement confrontés aux squatters vous savez si aujourd'hui, les copropriétés les copropriétés dégradées sont dans cet état-là, c'est parce que nous n'avons pas toujours eu tous les moyens de lutter contres les squatteurs. Si aujourd'hui la démolition du Chêne Pointu à près d'un an de retard, c'est parce que nous n'avons pas eu tous les moyens pour lutter contre les chasseurs, les squatters et vous le savez, comme élu du Val-de-Marne. Cette situation, vous la connaissez Madame Lienemann, vous êtes aussi. Actrice du logement social. vous ne permettait pas des des squatters de rester dans le logement social et vous avez raison de le faire parce que c'est insupportable d'avoir des squatters. Mais oui comme vous nous protégeons les gens en situation d'impayés de loyers. Oui comme vous et et je, j'y suis 13 attentif. Nous luttons contre les expulsions locatives parce que chaque expulsion locative est un échec et je continuerai à le faire, j'ai présidé depuis que je suis ministre toutes les CAPEX et tous les lieux dans lesquels nous travaillons pour les expulsions. J'ai réuni dernièrement l'ensemble des énergéticiens pour qu'ils mettent plus encore au pot du FSL parce que c'est leur devoir de mettre au pot du FSL et et pour ma part je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de leçons à recevoir. Merci. Merci Madame Lienemann pour explication de vote à verticale. Oui, chers. On nous répète à juste titre, quelques cas. Qui sont dramatiques, qui sont une personne qui voit son domicile. Habituel occupé par des squatters. Normalement, la loi protège déjà. Je ne sais que par quel incurie du système. On n'arrive pas à faire appliquer ce qui déjà est interdit car c'est évidemment interdit à la installé dans un logement de quelqu'un. J'aurais été tout à fait favorable à ce qu'on nous explique pourquoi la loi était mal foutu et qu'il fallait la durcir. Sur ce point. Deuxièmement tous les squats ne sont pas ça. Tout ceux effectivement qui sont du domicile. Et d'ailleurs Monsieur le Préfet, Monsieur, pardon, excusez-moi parce que. Saisie de temps en temps le préfet là-dessus monsieur le garde des Sceaux je vous enverrai la liste d'un certain nombre de bailleurs sociaux qui saisissent le procureur de la République pour des squats illicite de leurs locaux. De logements de logements sociaux. Classée sans suite systématique. Bon, mais pas son. sait pas, il y a des squats, qui sont des locaux vides depuis des lustres occupé. Par des squatters c'est pas bien, c'est sûr. Mais si ils sont pas là ils sont vous. Ça c'est la question que vous posez pas. Ils seront ou. Avec leurs gamins. Parce que je vous parle de pas de ceux qui occupent le domicile. Ils sont infimes. Mais cela vous pleurez pas sur leurs gosses. Qui vont être ou. S'ils sont pas là, la plupart du temps. La plupart du temps. Il y a pas assez de logements sociaux pour loger tous ces gens-là, vous le savez bien. Tous les maires le savent. Donc déjà on aurait pu être beaucoup plus pragmatique pragmatique et d'ailleurs je me rappelle le débat avec Madame Procaccia qui parlait bien du logement. Où vivaient les gens.

je pense que vous à d'autres moments vous aurez à vous exprimer, vous avez 2 minutes et je donnerai pas plus. Merci de respecter le règlement. Comme ma collègue, nous ne considérons qu'il n'y a pas lieu de légiférer à nouveau sur la question du squat. Bien évidemment que nous sommes tous ici contre l'occupation illicite de logements par des squatters. Avec la loi ASAP de 2020, le délai d'évacuation d'un squatteur est désormais de 72 heures, cela permet de mettre normalement de mettre fin rapidement aux occupation illicite de logement je ne sais pas pourquoi, moi non plus. La loi ne s'applique pas comme elle devrait s'appliquer et de plus depuis le 1er février 2022, un accompagnement et proposé aux propriétaires victimes de squat jusqu'à la restitution de leur logement. Il n'y a pas lieu de légiférer pour des mesures toujours plus répressives sans. Cacité supplémentaires, les petits propriétaires ne seront pas davantage protégés. S'agissant du 2ème volet de la proposition de loi qui est une atteinte aux procédures de prévention des impayés des expulsions locatives. Il n'y a pas lieu de délibérer non plus dans un pays qui compte 15 millions de familles fragilisées par la crise du logement dans un pays où le logement pour être la bombe sociale de demain. Comme vous l'avez si bien rappelé, Monsieur le Ministre du Logement ce texte hein dépanne texte de justice sociale. Contrairement à la présentation qui en est faite par la majorité présidentielle. Ce texte n'est pas équilibré car il accroît la pression sur les plus vulnérables de nos concitoyens, contrairement à ce que vous soutenez Monsieur le Ministre du logement en fait. Ce texte n'est pas du tout consensuel les instances de défense des droits de l'homme y sont fortement opposés ainsi que l'ensemble des acteurs de la solidarité et les services sociaux. En conséquence, notre groupe votera la question préalable déposée par nos collègues du groupe CRCE. Merci, cher collègue, Monsieur Bonhomme. Je ne vois pas en quoi le risque d'exclusion ou même de d'atteinte à la vie privée il viendrait tout justifier, y compris et les violations caractérisées de domicile. Et encore une fois et encore une fois nié complètement toute début de d'application du droit de propriété. Je voudrais juste faire une piqûre de rappel, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Non pas sur la déclaration Norodom de 1789 mais sur la constitution des 793. Qui a été validé, vous le savez. Par un certain Robespierre d'inconnus pour. Bien connu pour son sens de la mesure et son humanisme et. Dans l'article de la Constitution en réaffirmer le caractère sacré et inaliénable de droits de propriété et si c'était pas suffisant. Mardi 19, nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété propriété sans son consentement. Je crois que ça vaut tous les discours. Merci cher collègue. Monsieur le président Gontard. merci madame la présidente. Moi je voulais. Donner raison à à Madame Boyer qui s'est exprimé tout à l'heure. Oui effectivement il faut tout faire pour protéger nos concitoyennes et nos concitoyens. Je suis d'accord avec vous je voudrais rappeler un certain nombre de chiffre qui ont été cités ici parce que derrière ces chiffres Baya justement des femmes et des hommes qu'il faut protéger le nombre de personnes sans domicile dans son domicile fixe a été multiplié par 2 en 10 ans, on est à 330.000 aujourd'hui les chiffres. Des chiffres de la Fondation Abbé Pierre, 85.000 foyers reconnus au titre du DAL en attente de logement. 2 millions de demandeurs de logements sociaux, 4 millions de mal-logés, 3,1 millions de logements vacants. pardon, la rue a tué 623 personnes. Donc oui nous devons projet protéger nos concitoyens et nos concitoyennes le 115 ça a été dit refuse un hébergement à plus de 6000 personnes dont 1700 enfants, 42.000 enfants sont encore à la rue et sont sans abri en France. Est-ce qu'on peut se satisfaire de de ça, un logement sur 10 est vacant et c'est une hausse de 55% en 20 ans. les squats dont on parle c'est zéro 0. 0 5% des logements recensés donc je pense qu'on pourrait avoir peut-être reprendre un sens des des réalités que notamment le ministre du Logement, qui s'est exprimé et qui disait qu'il n'avait pas de leçon à recevoir, au lieu qu'on parle de de problématiques dont on sait que elles sont déjà puni par la loi et qu'effectivement il y a une question d'application de la loi qu'on parle par exemple ce soir de garantie universelle des loyers d'encadrement des loyers. De revalorisation des APL, ça on pourrait également parler de respect de la loi SRU ça également c'est quelque chose sur lequel on on pourrait parler et je pense que c'est des vraies solutions effectivement pour prendre de protéger nos concitoyens et nos concitoyennes si. Je rappelle que c'est une expression par groupe politique. Merci. Alors je vais consulter le Sénat sur la motion tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte, en discussion j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste solidarité et territoires sur la motion numéro 6 tendant à opposer la question préalable. Je vous rappelle que l'avis de la commission et du Gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Le résultat du du scrutin nombre de votants 344 exprimés, 344 pour 91 contre 253 le. C'est n'a, n'a pas s'adopté. dans la suite de la discussion générale. La parole est à monsieur Denis Bois-d'pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 9 minutes, chers collègues. Madame la présidente, messieurs les ministres. Madame, monsieur le rapporteur, chers collègues. Bien souvent, pour être pertinente et efficace. Une mesure politique doit s'inscrire dans une langue timing. Et porter un juste équilibre. Ce texte, sur lequel autres assemblées de débattre aujourd'hui ne satisfait pas ces 2 exigences. À mes yeux il est ni équilibrée ni dans la bande de temporalité. Sur un sujet comme celui-ci, la complexité relève de l'arbitrage. Entre le droit à la propriété et le droit au logement. Concrètement, il s'agit de concilier la protection des locataires et celle des bailleurs. Nous nous demandent de faire la différence entre certains faits divers. Dont on a beaucoup parlé. Et divers médiatisés la réalité des chiffres qui nous démontre que, fort heureusement. Ces situations reste exceptionnel. Dans son rapport, le défenseur des droits, indique d'ailleurs que le squat reste un phénomène très marginal. En 2021. Sur l'ensemble du pays. Seulement 160 squat. De domicile aurait été signalé. Selon les chiffres communiqués par le rapporteur par le rapporteur de survie. Il y a eu environ que 40 cas d'intervention effective de la force publique. Dans une grande majorité des cas les propriétaires ont pu retrouver leur logement. Ça nous a passé par la justice. La loi d'accélération et de simplification. De l'action publique, adoptée en 2000 ovins a également permis d'accélérer les procédures liées à l'occupation illégale dans le logement. Cela témoigne notre arsenal législatif actuel. Qui nous permet d'adjoint d'apporter des réponses à ces situations. Aussi sur ce point ne tout trouvant assez bien dans la position du président de notre assemblée. Qui, lors de ses voeux. Appelé à une certaine forme de sobriété législative. Plutôt que de légiférer. Une nouvelle fois sur ce sujet. Veillant à l'application du droit existant. Au-delà de la simple question du quoi. La protection des propriétés. Les situations abusives et tu pris refuge patients plus que légitime. Nous devons la traiter tout en conservant l'ambition de limiter les expulsions qu'en cas de dernier recours. Celles-ci sont bien sûr parfois nécessaire. Pour libérer le bien d'un propriétaire. Mais ça ne reste pas moins des situations humaines qui sont derrière compliquer. La réduction des délais de paiement des contentieux telle que prévue dans cette programmation de loi Robien code tout le travail d'accompagnement social et de relogement. C'est d'abord la question de l'efficacité. Dans des délais aussi contraints. Comment mobiliser les à de nécessaires à la régularisation de la dette.

Prévoyait de limiter ce délai à un mois. Madame et messieurs les rapporteurs. Vous avez reconnu le caractère contre-productif de réduction de la période au cours de laquelle la majeure partie des impayés se résolvent. Vous avez un ramener ainsi le délai à six semaines.

Donc concrètement, mes chers collègues. Ce texte nous ramène à légiférer sur les réduire les délais de procédures de prévention aux élus, aux aux expulsions de deux semaines en y revient. C'est parfait. Au-delà de l'efficacité de ce mesure l'entendent peut douter. Est-ce que collectivement d'entre gens c'est notre priorité dans le pays où les difficultés d'accès et le maintien dans leur logement persistent, voire s'aggravent. Avec mon groupe, nous demandons le mêler le maintien du délai actuel nécessaires pour prévenir les expulsions. Trouver les solutions de reprise de paiement. Et au besoin et mettre en place. Un accompagnement social. Il s'agit là d'une demande forte. Et l'ensemble des acteurs de la solidarité. Je tiens néanmoins à reconnaître le travail de la rapporteure qui a permis de supprimer certaines dispositions totalement déraisonnable qui aurait été dans le croit dans le texte de loi et qui aurait été transmise par l'Assemblée nationale. Je pense à l'amalgame qui est fait entre squatteurs. Et locataires locataire un défaut de paiement. Je pense aussi à la suppression de certaines prérogatives que le juge. Peut exercer d'office et dont il est question de conditionner la demain à la demande des locataires. Cela traduit l'ambition des auteurs de ce texte qui de déséquilibrer le système existant en fragilisant les locataires en difficulté et souvent de bonne foi. Je salue également la proposition de renforcer le rôle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. Mais, mais qu'en sera-t-il des moyens concrets pour agir. Y aura-t-il davantage de personnel pour accompagner cette évolution. Si pour les raisons que je viens d'évoquer le contenu de cette proposition de la de loi nous pose question. Toujours interrogé aussi sur la temporalité. Dans cet hémicycle, nous avons régulièrement l'occasion de débattre sur la crise du logement qui traverse notre pays, il y a quelques semaines seulement lors de l'examen de projets de loi sur les finances. Nous étions nombreux sur les différents bancs de cette assemblée à partager cette préoccupation. Aujourd'hui en France. 14. Plus de 6 millions de personnes. Fragilisée par la crise du logement. Plus de 4 millions sont mal logées. 300.000 sont sans domicile. fois des foyers sont en situation de précarité énergétique. De de de. Il y a 2 le demi million de ménages sont en attente d'un logement social. Face à cette crise du logement. Cette proposition de loi est à contre-emploi et à. Nous savons Nous savons qu'il existe des propriétaires qui peuvent se retrouver eux-mêmes dans une situation difficile. Car ils subissent les impayés de loyer de la part de leurs locataires. Ces situations ne sont pas acceptables. Nous devons les regarder en face et bien sûr nous devons y répondre.

Elle-t-il de nature à insister. Les investissements locatifs. Est-il de nature à alléger les procédures de sélection rappliquer au moment de la mise en en location. Monsieur le Ministre. Les rapports entre propriétaires et locataires sont importants. Mais la réalité, la réalité c'est qu'aujourd'hui. Que ce soit pour l'occasion l'achat les logements sont de plus en plus accessible à une grande partie de nos citoyens.

En réponse à l'explosion des dépenses de logement. Nous devons réfléchir à une réévalue uberisation des aides au logement. Et notamment la Real l'avait a eu évaluation du forfait charge des APL. Nous devons agir sur le prix du. Si un État à Bruno et à la stratégie de mobilisation du foncier public. Nous devons également permettre une réappropriation du bâti existant à travers un grand plan de rénovation afin de lutter contre la vacance qui impacte un 1er lieu les territoires ruraux. Je rappelle à ce triste ce titre que plus de 3 millions de logements sont actuellement vacants. Bien sûr nous devons légalement accroître nos efforts en matière de rénovation énergétique un de favoriser la rénovation globale qui ont une réelle incidence sur la facture énergétique. Enfin. Nous devons construire. Plus de logements sociaux, la fragilisation financière des acteurs à enrayer la dynamique de construction de ces dernières années. Nous devons impérativement trouver un nouvel élan. Monsieur le Ministre, à vous disiez 125.000 logements par an 250 omis de ce logement sur deux à nous en sommes à peine à 85.000. Alors alors qu'il était député.

Messieurs les Ministres, chers collègues à reprenant cette géologique. Comment sécuriser les propriétaires bailleurs sans se préoccuper des locataires en difficulté des politiques volontaristes visant à diminuer le poids des dépenses de logement dans le reste à vivre. Les Français ne sentaient le pas la meilleure garantie que l'on peut apporter aux petits propriétaires. Au sein du groupe sénateur socialiste pensant que nos politiques ont tout à gagner en termes d'efficacité lorsqu'elle s'attaque aux causes plutôt que de traiter les symptômes. Si, si certains amendements qui sortent du bâtiment dans le bon sens. Merci. Nous sommes la Madame la présidente. Monsieur le Ministre. mes chers collègues, je vais d'abord. Peut à tout le monde ici je ne convoquerait ni Robespierre ni Jean Jaurès mais plutôt parce que l'urgence est là. Les 400 millions de mal logés les 170 propriétaires spoliés pour rappeler ici que ça te PPL ne règle rien et ne répond en rien au problème crucial de notre pays, celui d'avoir un logement digne et les périodes récentes de confinement ont démontré l'importance de la qualité d'un logement pour bien vivre. Alors vous nous proposez une PPL qui porte un coup violent au progrès collectif pour prévenir les expulsions locatives et les mises à la rue. De fait, elle fait fi des plus précaires. Sous couvert de rééquilibrer les rapports entre locataires et propriétaires. Vous nous proposez de criminaliser la précarité.

Et d'ailleurs le droit actuellement en vigueur est insuffisant pour y répondre. Mais l'objet de cette proposition de loi n'est donc pas de résoudre cette situation. Au contraire elle stigmatise les plus pauvres, ces femmes, ces hommes qui locataires n'ont pas les moyens de payer leur loyer dans des zones où la spéculation le profit rendent le loyer de plus en plus cher ou les locataires sont de fait précarisée et où le nombre de SDF ne cesse d'augmenter. À l'inverse nous réaffirmons qu'aujourd'hui l'urgence est de défendre le droit au logement, le droit de chacun à une vie digne, quelles que soient ses difficultés, l'urgence est d'éviter que davantage de personnes et de familles en situation de précarité ne se retrouve demain à la rue. Criminaliser aujourd'hui la précarité sans même un mot contre les bailleurs spéculateurs et autres marchands de sommeil qui empêchent l'accès à un logement abordable stable et décent plus pauvres est inacceptable dans une République qui arbore avec raison sa devise Liberté, égalité, fraternité sur les frontons de toutes nos mairies. Concrètement, ce texte prévoit une accélération considérable de l'expulsion des locataires en impayés de loyers, empêchant tout travail sérieux d'accompagnement et retirant à la justice, son pouvoir d'appréciation. Actuellement, ce sont environ 300.000 personnes qui sont sans domicile plusieurs millions de personnes mal, voire très mal logés dans un pays qui regorge de plus de 3,1 millions de logements vides. La plupart de ces personnes occupent pourtant un emploi souvent précaires qui ne leur permet pas d'assumer l'ensemble des dépenses. Aucune de ces personnes ne s'invite chez l'autre pour pouvoir y passer une nuit tranquille. Ainsi, à l'heure de voter ce texte. Ayons conscience qu'une personne expulsée ne pourra pas trouvé d'hébergement des familles à la rue et donc encore moins un logement. Elle est condamnée à vivre dehors et ceux éventuellement avec sa famille. Alors Monsieur le ministre et le représentant de la majorité présidentielle. Vous pourriez me répondent que certes c'est une réalité mais qu'il ne revient pas aux propriétaires de faire les frais de la pauvreté de plus en plus importante pour nombre de nos concitoyens. Je vous répondrai alors. Mais que fait le gouvernement, que fait la majorité présidentielle pour la résorber. Où sont les nombreuses propositions de loi pour permettre de s'attaquer résolument à à la spéculation foncière et immobilière qui rendent de plus en plus inaccessible. L'accès au logement dans les grandes métropoles, là même où le travail précaire se concentre. Que fait la majorité présidentielle pour assurer des salaires et des pensions digne qui permettent de pouvoir se loger sans avoir à arbitrer. En début ou le ou le 15 du mois. Entre payer son loyer, sa facture d'énergie remplir son frigo ou satisfaire aux dépenses de l'éducation de ses enfants. Alors la facilité qui visent à stigmatiser le plus démunis n'est pas acceptable et dans notre groupe, nous l'avons toujours refusé. C'est d'ailleurs à l'inverse un tout autre projet que nous souhaitons pour notre pays. Nous ne pouvons donc ici ce soir que dénoncer une telle proposition de loi qui in fine et et au vu des premiers débats que nous avons eu parfois un peu chaotique ici au Sénat ne sert finalement ni les intérêts des propriétaires ni ceux des locataires et en l'état, bien évidemment, vous l'aurez compris, notre groupe votera contre sa proposition de loi. Merci, cher collègue, la parole est à madame Nathalie Goulet, pour le groupe Union centriste et pour quatre minutes. minutes. Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Mes, mes chers collègues. Madame la rapporteure Estrosi Sassone. À cette heure tardive, beaucoup de choses ont été dites dans le cadre d'émotions qui aurité. Présenté et défendu et et je dois dire que j'ai un certain malaise avec ce texte et le manichéisme qui qui ressortent de nos débats, il y aurait les gentils qui voudrait protéger les mal logés, et puis les méchants qui voudraient protéger les propriétaires là ne justifiant pas l'autre et vous l'avez dit, Madame, Tucker mal c'est pas parce qu'on est mal logé, qu'on doit aller squatter l'appartement de de quelqu'un d'autre. Donc ce débat à une heure tardive comme je viens de le dire, laisse une une une espèce de de saveur un peu un peu douceâtre et en tous les cas. Une odeur de de manichéisme qui me semble mal adapté le texte, je vous le rappelle le porte sur l'occupation illicite des logements et pas sur l'ensemble de la la politique du logement, on l'a dit 500.000 comment commandement de payer 160. 15.000 expulsions. Des propriétaires qui sont évidemment lésés et notamment des retraités qui ne peuvent pas toucher les loyers qui leur permettrait d'améliorer leur retraite, et également des propriétaires des propriétaires qui hésitent à mettre des appartements en location de peur évidemment de ne pas être payé de leur loyer. Alors de ce point de vue là, je voudrais rendre hommage à nos 2 rapporteur André Reichardt et et Dominique Estrosi Sassone virtuose. Du sujet avec Valérie Létard et Marie-Noëlle Lienemann qui sont dans cette maison, les grands spécialistes. Du logement car vous avez les uns et les autres et le travail de notre commission a complètement rééquilibré ce texte et effectivement le texte fait tout à fait la différence entre des. Locataires qui ne payent pas leur loyer et et des squatters sans droit ni titre le le texte de la commission de ce point de vue est absolument clair et je ne crois pas qu'il y ait du tout d'amalgame entre les deux. Donc, notre groupe soutiendra le texte tel qu'il ressort de la rédaction de notre commission. Le cap doit être fixé d'une loi utile et équilibrée. Une loi utile parce qu'elle doit envoyer un signal clair aux squatters et aux locataires abusive et se traduire par des effets visibles sur le terrain. Plusieurs amendements adoptés comme je l'ai dit constitue évidemment un un apport une loi équilibrée ensuite dans l'objectif de mieux sécuriser les rapports locatifs, on discute en distinguant clairement clairement la situation du squatteur de celle du locataire, accumulant les impayés. C'est ce que je viens de dire. Mais j'avais précédé mes notes. Nous avons en commission souhaitait également conserver la possibilité pour le juge d'accorder des délais à locataire faisant l'objet d'une décision d'expulsion et je crois qu'il y aura aussi des amendements dans ce sens sens qui seront présentés en séance parce qu'il faut aussi laisser aux locataires en difficulté la possibilité. De rattraper ses loyers impayés sans l'entraîner dans une spirale de l'exclusion qui, nous le savons les uns et les autres est une spirale. Mortifère. Notre objectif est donc clairement de lutter contre la violation du droit de propriété que constitue le squat. Nous souhaitons pas mettre en difficulté les locataires de de bonne foi. C'est en alliant ses considérations d'efficacité de justice que nous parviendrons à rétablir la confiance des Français dans la propriété et la confiance des propriétaires dans la location c'est donc sous ses bénéfices de ces observations que notre groupe votera ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il est aujourd'hui une aberration, une injustice dans notre droit qui rend moins condamnable squatteur pénétrant un logement qui ne lui appartient pas que le propriétaire en expulsant par ses propres moyens où où le squatteur encourt un an de prison et 15.000 euros d'amende. Le propriétaire lui encourt 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende. Il y a un problème avec le droit de propriété dans notre pays. C'est pourtant quasiment le 1er droit constitutionnel après la liberté. Il serait temps d'y mettre fin. Car encore en 2019, le député la glaise a remis à la demande d'Édouard Philippe, un rapport indiquant je cite que le foncier même propriété privée demeure un bien public fini et d'intérêt général. Une véritable remise en cause des fondements de notre contrat social par la majorité macroniste au pouvoir. De son côté, la gauche, 33 ans après la chute du mur de Berlin promeut encore la collectivisation des propriétés privées, sauf les siennes bien entendu et entretient une anachronique lutte des classes entre locataires et propriétaires quitte à faire de l'électoralisme sur l'anarchie ambiante. grand coeur mais vous oubliez que la majorité des propriétaires sont de petits propriétaires et que leur vient est le fruit d'une vie de labeur qu'souhaitent légitimement protéger pour en obtenir un complément de retraite et transmettre à leurs enfants plutôt que de le voir occupé et saccagé par des marginaux ou des migrants. Vous avez grand coeur mais vous oubliez que la plupart des squats sont le fait de clandestins ou de mafias étrangères problème que vous avez largement contribué à importer. Vous avez grand coeur mais pas assez grand pour y accueillir ce couple de retraités marseillais condamné à vivre sur un Parking pendant 2 ans et demi après avoir trouvé après avoir travaillé toute sa vie et ce en raison du squat de leur appartement vous en appeler à la solidarité à une sous la solidarité sélective toujours en fonction des squatters jamais en direction des propriétaires lésés. Mais que se lève dans cet hémicycle dans cet hémicycle il y a sept à sa gauche, en particulier les volontaires qui accepteraient de vivre au nom de la solidarité. Le squat de leur de leur logement ou de leur résidence secondaire. A choisi entre le camp de l'incitation au squat et celui de la sanction. Je suis du côté des seconds mais je rajouterais tout de même qu'on ne fait aucune bonne politique en s'attaquant aux seules, conséquence d'un problème surtout quand on enchéri les causes. Le 10 mai 2022 CIV migrants ont été évacués de 34 logements dans trois bâtiments différents dans la cité du parc disent à Marseille les squats de Roms à Marseille se multiplient, avec le soutien de la de la municipalité d'extrême gauche plurielle qui envisage même de crier, de créer un village rom l'immigration anarchique participe activement activement à la hausse de ce fléau grandissant. La propriété est une ZAD une zone à défendre Jean Seri ici au nom de la justice et des droits des honnêtes gens. L'un des défenseurs. Merci cher collègue. La parole est à monsieur. Jean-Yves Roux pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes. Madame la présidente, messieurs les Ministres Madame et messieurs les rapporteurs chers collègues lorsque nous examinons les textes alors du jour de notre chambre haute. Nous pouvons difficilement les sortir des contextes économiques et sociaux que nous traversons. En effet, cela a été maintes fois évoquée depuis la fin de l'année 2021 et encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine, les particuliers subissent de plein fouet l'envol des l'indice des prix à la consommation, en particulier sur les dépenses énergétiques. Malgré un bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, la remise à la pompe pour le carburant le chèque inflation, les difficultés internes du pouvoir d'achat perdure impact hein de fait la répartition et le niveau des dépenses de consommation des ménages français. Cette progression de la précarité financière s'observe au quotidien. Notamment à travers l'intensité des actions des associations de solidarité, sur le terrain. Ces données centrale nous ont dans un 1er temps fait penser que cette proposition de loi visant à protéger les logements montres l'occupation illicite semblé quelque peu anachronique un miroir avait l'urgence sociale. Nous nous étions donc pas pleinement en phase avec l'identification de la cause afin de traiter le problème à sa source. Pour autant, les quelques rares affaires de squat qui ont été médiatisés ne nous laisse pas indifférent. Nous sommes parfaitement conscients du trouble que cela représente pour le propriétaire car la détention de bien suscite la plupart du temps, un sentiment de fierté et d'accomplissement. Ainsi les mois d'un propriétaire en face à une occupation illicite était et compréhensible, qui plus est lorsqu'il est alimenté par une impression d'impuissance par conséquent pour éviter de glisser dangereusement vers des situations où où les propriétaires feraient justice eux-mêmes avec les pires scénarii que l'on peut imaginer légiférer Sam d'une voie rationnelle de surcroît lorsqu'il existe vraisemblablement une volonté politique partagée de légiférer. Un but d'améliorer le cadre juridique dans ce domaine en effet en dénombre pas moins de 20, proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale et au Sénat depuis 2020. Vous l'aurez compris, nous ne m'ils n'auront pas ces sujets de contentieux locatif mais nous restons vigilants pour que cela ne donne pas lieu à des reculs significatifs sur le droit au logement. Notre groupe a donc formulé des demain vise à infléchir un texte qui déséquilibre peu ou prou les rapports propriétaire locataire. Nous défendons notamment que l'information selon laquelle les locataires en seule la faculté de demander au juge de leur accorder les délais de paiement soit bien connu des locataires concernés. Par ailleurs, nous nous opposons à la réduction des délais entre le commande demain à payer et la résiliation automatique de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement. Les tensions du marché locatif et les difficultés à trouver une solution de relogement aux locataires rencontrant des difficultés financières sont trop fortes pour mettre à mal l'accompagnement social pratiqué dans l'intervalle. Nous faisons aussi le pari d'un dialogue et d'une négociation amiable entre le locataire et le bailleur sur la surveillance d'un commissaire de justice. Ses contributions aux articles 4 et 5 sont de nature à compenser des asymétries d'information dans les locataires. On peut en faire face. Un cas de contentieux. Mais nous partageons en revanche l'inquiétude des associations de solidarité à l'image de la Croix-Rouge et du Secours catholique ou de la Fondation Abbé Pierre, sur la question de la pénalisation des locataires qui se maintiennent à leur logement a pris une décision définitive de justice. Le propriétaire bailleur ne doit pas se situer à l'état dans son rôle d'accès au logement garanti dans l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Enfin toujours dans un souci de compenser la rigidité de cette PPL il serait opportun de renforcer le budget consacré à l'hébergement d'urgence au moyen pour les équipes mobiles et les a que deux jours. En conclusion, le groupe RDSE est pleinement mobilisé pour avancer sur ces sujets et il regrette l'aspect équivoque d'une proposition de loi qui fait l'amalgame entre l'occupation illicite et les impayés de loyers. Par respect pour notre tradition et la diversité de nos opinions nous appliquerons notre principe de liberté de vote sur le texte à se partageant entre le pour et l'abstention. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Stéphane Le Rudulier. Pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

Madame la présidente. Messieurs les les ministres ce président de la commission des lois. Madame la rapporteure chers Dominique monsieur le rapporteur. André, mes chers collègues. Effectivement. Maryse et Pierre, ça a été cité, c'est un exemple parmi tant d'autres ont récupéré il y a quelques semaines de cela après plus de 2 ans de de combat. Leur leur logement qui était. Occupé illégalement par une. Une individus qui a enfin quitté les lieux après. L'intervention des des forces de l'ordre. Mais des cas comme. Maryse et Pierre il en existe des centaines dans notre pays. J'aurais pu. Citer l'exemple également de Marie-, Thérèse et et Henri. Des personnes retraitées de Théoule sur Mer. Aurait été désespéré au vu du saccage de leur domicile après. 30 années de dur labeur d'économie pour devenir propriétaire en fait ce sont et c'est de cela dont il s'agit des des honnêtes. Citoyens qui sont privés de leurs maisons privées de de leur appartement par. Des squatters et ces honnêtes gens sont contraints de dormir ailleurs donc parfois dans leur voiture, parfois même. Dans la rue. Et ne nous y trompons pas, ces, ces personnes qui s'approprie. Des propriétés privées par effraction. Ce ne sont pas des des Robins des Bois. Des temps modernes. Il n'existe aucun romantisme au vol. Et n'ayons pas peur. Des mots. Ces squatters font des délinquants qui veulent le bien le plus intime. D'une famille à savoir. Le foyer. Et le squat, c'est en quelque sorte. Permettez-moi ce ce parallèle. Un cambriolage. Ou le voleur. Reste. Dans votre salon. Et s'y installe. Pour y vivre les pieds sur la table. Et aujourd'hui, ça a été dit d'ailleurs par plusieurs d'entre nous, c'est un véritable système organisé de squat qui se met en place, profitant des failles de notre droit aujourd'hui. Ça a été souligné. Monsieur le Ministre la rappeler. Il y a même des guides. Sur Internet. Qui. Permet qui explique comment récupérer. Repéré le bon logement Le Bon propriétaire qui explique comment maintenir la police à distance. Ou encore comment pirater un circuit savoir si l'eau ou l'électricité sont bel et bien coupés. Et effectivement. Pour lutter contre ces squats les dispositifs existants, notamment la loi Dalo en matière de de répression, de fait de squats ne sont ni suffisamment dissuasif à l'égard des squatters ni suffisamment connu. Des préfectures, des forces de police ou de gendarmerie. Voir des propriétaires eux-mêmes le résultat nous le connaissons. C'est parfois l'incompréhension, le désarroi de propriétaires. Privés de leurs biens pendant des mois voire des années, qui ont véritablement l'impression que l'État respecte davantage les squatteurs que le droit de propriété. la République doit être toujours du côté de la justice et donc des propriétaires qui sont les victimes de ces situations indignes et en disant cela, il n'est pas question pour nous d'ignorer certaines situations désespérées de locataires qui n'arrivent plus à honorer leurs loyers. C'est une situation totalement différente et. En ce sens, le texte issu de la commission. Il me paraît très équilibré quand il appelle à la fermeté. Et à l'action contre le squat mais également une certaine forme d'humanité notamment par une sécurisation accrue des rapports locatifs ou par un meilleur accompagnement également des locataires en difficultés, notamment financières. Mes chers collègues. Ça a été dit par. Mon collègue. Bonhomme effectivement. Il y a eu la nuit du 4 août 1789. Après la prise de la Bastille. Qui symbolise la fin de l'ancien régime. il y a eu l'abolition de la la féodalité et l'Assemblée nationale constituante. Cette nuit-là a posé les fondements de notre conception contemporaine de la propriété individuelle et privée forcément privés et. Mes chers collègues, clairement il s'agit ici dans cette PPL de préserver le droit au logement. Nous devons avant tout préserver le droit à la protection de la propriété immobilière. C'est tout l'objet de ce texte durcissant les peines pour ceux qui viole le domicile d'autrui sanctionnons tout acte de propagande et publicité en faveur des méthodes visant à faciliter ont incité les squats et donnons les moyens au maire et à l'État d'agir rapidement.

Madame la présidente. Monsieur le garde des sceaux. Madame, madame, monsieur le rapporteur. J'avais un propos qui était prévu, mais comme il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je vais éviter au maximum au maximum les redites et puis j'ai pris des notes au fur et à mesure des, des débats qui ont été tenus et j'espère que mon propos sera que Pour dire à certains collègues qu'il y ait des tensions très fortes sur le logement social sur les territoires. C'est vrai. Qu'il faille lutter et chacun de nous le faisions quand nous étions mer ou en responsabilité locale. Lutter contre le logement vacant. Bien sûr qu'il y ait des difficultés de mal-logement. C'est évident. Qu'il faille lutter contre contre les marchands de sommeil, qu'on a tous connu aussi dans nos communes. Sur le thème je vois bien qui respecte assez peu de choses je touche les APL par la CAF en Direct sur les comptes et je ne m'occupe pas du propriétaire qu'il faille lutter con tout ça oui oui oui. Sauf que c'est pas l'objet de ce texte en fait. Cette proposition de loi, elle s'appelle protéger enfin elle vise à protéger les logements contre l'occupation illicite. Et sont concernés évidemment des professionnels des bailleurs mais ça a été dit, une immense majorité qui sont des propriétaires qui ont un bien. Des fois deux, des fois trois et c'est pas un drame, ça s'appelle la propriété privée, ça s'appelle le capital-, ça s'appelle bâtir un Patrimoine.

et les dispositions d'équilibres qui sont apportées dans ce texte dans un 1er temps, la proposition sanctionne plus durement les intrusions et les plus que les occupations illégales des domicile. Face au développement de ces pratiques, il était nécessaire d'envoyer un message de fermeté. Le droit de propriété doit être respectée. Cela ne vaut pas seulement pour les domiciles mais plus généralement pour tous les immeubles qu'ils soient usage économique ou à usage d'habitation. Nous saluons donc l'aggravation des peines des infractions concernées. Si vous me permettez un mot comme beaucoup ont abordé le sujet sur les squats et je ne parle pas forcément du squat dans le domicile des gens qui habitent. C'est, c'est totalement inacceptable. Je parlais du squat dans un logement qui appartiendra quelqu'un qui est vacante temporairement. Il est choquant de voir des associations jusqu'au-boutiste des représentants des élus parfois alors c'est pas c'est pas ce que j'ai entendu ici mais le dernièrement j'ai entendu la maire de Nantes soutenir ce type. De démarche. j'aimerais quand même voir leur réaction. Si elle-même propriétaires de logements dans lesquels il y avait rien ni personne. On venait de l'occuper. J'aimerais voir comment on passe de la théorie à la pratique. Je serais assez assez curieux de voir notre chère collègue qui s'est exprimé tout à l'heure madame la la mais la ministre. Vous preniez l'argument de dire. Posez-vous la question de pourquoi des gens vont dans des squats. Mais si on démarre comme ça mais comment on bâtit une société. je veux dire, si vous trouvez une excuse une fois pour des gens qui occupe illégalement un squat. Vous mettez le doigt dans un engrenage dont vous ne sortez plus une société se bâtit avec des règles avec un cadre et après une capacité qu'on se donne à faire appliquer ces règles et ce cave ce texte, c'est une bonne chose puisqu'il raccourcit les délais de la procédure d'expulsion. Il n'est pas normal que les propriétaires hors période de trêve hivernale doivent en plus faire face à d'importants délais tout au long de son examen à la commission a souhaité à juste titre différencier le squatteur du locataire mauvais payeur. L'un est entré par effraction, l'autre pas. La commission des affaires économiques a également utilement enrichi le texte en améliorant le traitement des impayés locatifs avec une meilleure prévention et un meilleur accompagnement ces dispositions bénéficieront tantôt locataires, copropriétaires le groupe les indépendants votera en faveur de ce texte jugé utile et équilibrée et comme il nous reste un peu temps madame la présidente. Un mot sur l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, la fameuse ZAD. peut-être que le sujet est pas directement lié. Mais enfin si on s'entrave. À l'échelle des territoires pour ne plus pouvoir construire enfin je veux dire moi, il y aura de logements qui se construiront plus il y aura de tension sur le logement. Bon la police dirait pas mieux l'argument peut être pas très mais c'est des question qu'il va falloir qu'on se pose dans les semaines et les mois qui viennent mais que mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. La parole est à Monsieur Daniel Salmon pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour cinq minutes.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre. Madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Cette proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite constitue un grave recul du droit au logement sous couvert d'une volonté de protection des petits propriétaires. Le texte initial stigmatiser une population socialement précaire au lieu de créer les protections nécessaires, aussi bien pour les locataires que pour les bailleurs. Le texte issu de la commission n'à vrai dire guère meilleure et si limite quelques attaques contres les locataires en situation d'impayés. Il aggrave certains pans répressif du texte. Une loi d'affichage qui vise à monter en épingle. Quelques rares affaires de squats récemment médiatisé. L'Observatoire des squats n'a dénombré que 170 cas. Vous me direz c'est déjà beaucoup, mais 170 cas en 2021 et la majorité de ces cas ont été résolus. Si la propriété locative doit être protégé les violations de domicile sont des situations graves qui doivent être punis. J'insiste là-dessus. Encore une fois, elles sont exceptionnels et l'arsenal juridique permettant d'y mettre fin, existe. Et ce n'est pas par la stigmatisation et la Crimée criminalisation des locataires les plus précaires que nous pourrons mieux protéger ce que vous prétendez défendre. Face à la crise du logement et à la crise sociale qui s'aggrave de jour en jour. Vous n'avez donc rien trouvé de mieux. Que de faciliter les expulsions pourra payer de loyer criminaliser plus encore les occupants sans droit ni titre, comment imaginer a-t-elle. Retour en arrière, au moment où de plus en plus de familles sont précarisés par la hausse des prix des loyers de l'énergie et par l'inflation d'un bout à l'autre. Ce texte est unique inutile et dangereux. Le groupe écologiste s'opposera fermement à ces mesures notamment celles qui prévoit une peine totalement disproportionnée à l'encontre des occupants de logements vacants. Celle qu'il qualifie de vol l'occupation sans droit ni titre de tout local à usage d'habitation ou à usage économique. Cet article fait primer de manière absolue la propriété immobilière sur la nécessité pour une personne de disposer d'un logement. Si la commission a mis fin à l'amalgame entre squatteurs et locataire défaillant. Le texte concerne le délit consistant à ne pas s'auto-expulsé de son logement. Dans les faits, parce qu'il faut regarder les faits, cela signifie qu'une mère de famille avec ses enfants en situation de pauvreté et ne pouvant plus payer de loyer devrait les emmener dormir sous les ponts pour éviter la prison. Non vraiment un locataire en difficulté un mal logés n'est pas un délinquant. Nous nous opposerons à la criminalisation des associations et des groupes militants dont l'action essentielle aident à garantir les droits et les libertés des personnes en précarité ou sans logis. Nous dénonçons également l'extension de la notion de domicile à toutes les propriétés privées étendre à tout type d'habitations les dispositions applicables au domicile est une conception absolutiste du droit de propriété et met de côté le principe de dignité humaine, ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle qu'est le droit au logement. L'article 5, enfin qui réduit les délais durant lesquelles les locataires en difficulté peuvent régulariser leurs impayés est une mesure particulièrement contre-. Le délai entre l'assignation et l'audience servant à mettre en mouvement tout le processus de prévention de l'expulsion. Et donc du sans-abrisme il protège les intérêts des locataires et des propriétaires. Alors que la rue affecte gravement la santé physique et mentale et a tué 623 personnes en 2021. Alors que le 115 refuse chaque soir un hébergement à plus de 6000 personnes dont 1700 enfants. Faut-il vraiment punir d'une peine de prison ceux qui s'abritent eux et leurs familles dans un immeuble entièrement vide depuis des années. Cette proposition de loi ne répond aucunement aux vrais enjeux du logement d'aujourd'hui vous prétendez sécuriser les rapports entre les propriétaires, les bailleurs et les locataires. Mais vous ne vous attaquez pas aux problèmes à la racine. Le bilan du gouvernement en la matière ne plaide pas en sa faveur. Vous avez fait du logement social, le parent pauvre des politiques publiques émis grandement à mal les offices HLM vous avez baissé les aides au logement et économiser plus de 1,5 milliards d'euros par an sur le dos des allocataires et vous ne menacez maintenant des milliers de locataires en est payé du fait de la hausse constante des loyers du coût de la vie de la baisse des APL ou encore de l'insuffisance des logements sociaux. Il y a pourtant des alternatives pour concilier le droit au logement avec le droit de la propriété. Il est temps de mettre en place la garantie universelle des loyers qui permet un accès plus facile aux logements pour les locataires sécurise les propriétaires et prévient les expulsions, mettez en place, encadrement des loyers qui réduit les vacances de logement et permet aux propriétaires de trouver plus rapidement un locataire. Monsieur le Ministre, attaquez vous enfin à cette crise historique du logement plutôt qu'à ses victimes. Ainsi qu'aux 3,1 millions de logements vacants. Opposez-vous à cette proposition de loi qui est une terrible règle des questions sociales et démocratiques. Je vous remercie. Merci la parole est à monsieur. Président François Patriat pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour six minutes. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, madame et monsieur le rapporteur. Le groupe RDPI a souhaité inscrire à l'ordre du jour, l'examen de la proposition de loi de notre collègue député Guillaume Kasbarian. Visant à protéger des logements contre l'occupation illicite. Elle est examinée dans le prolongement de la loi de 2020 et du texte proposé par notre rapporteur en 2021. Elle permet d'une part de sanctionner davantage du squat qui n'est plus un phénomène marginal, mais aussi de répondre au problème de contentieux locatifs à long terme. C'est également un texte qui, fruit de plusieurs compromis à l'Assemblée nationale que nous avons souhaité inscrire au Sénat pour l'enrichir l'améliorer l'équilibrer pour mettre en avant ce sujet d'une extrême importance qui n'est plus un phénomène marginal, autant qu'il les locaux. Nous avons quasiment tous été confronté à cette situation un administré petits propriétaires qui aura acheté un appartement à la sueur de son front ou un héritier d'une petite maison familiale retrouvons à bien ce face à ces procédures longues à des procédures longues qui peuvent durer jusqu'à 3 ans il y a des pseudos connaisseurs du droit au logement n'hésitant pas à narguer leurs victimes. Les propriétaires se retrouvent souvent démunis en grande précarité dans une profonde détresse psychologique, que ce soit en Île-de-France dans les Hauts-de-France ont Guyane Ont d'ailleurs reçu 200 témoignages et ont pu auditionner des 10 victimes dans les récits sont insupportables. Chers collègues, non le droit au logement n'est pas le droit au squat. Ce que nous affirmons clairement au sein du 1er chapitre de cette proposition de loi, c'est le squat doit être sévèrement puni. L'article 1er et promis en témoigne avec notamment un alourdissement de la peine encourue en cas de violation du domicile tout en évitant l'amalgame entre squatteurs et locataire défaillant. Et je tiens, ici, à remercier le travail des rapporteurs qui ont mené ce rééquilibrage sans tomber dans les travers idéologique ou dogmatique pour bien distinguer les squatters qui entrent illégalement dans un domicile de celui du locataire qui rencontrent des difficultés pour payer son loyer. Il en est de même pour l'incitation au squat dorénavant cette propre cette propagande soit sanctionné d'une amende de 3750 euros. Quel que soit le mode de plus, le texte que nous examinons il à sanctionner les abus et les escroqueries de faux propriétaires ils ne resteront pas plus impunis quand nous relevons le quantum de la petite de la peine prévue au sein du code pénal en les condamnant à 3 ans d'emprisonnement. Il y a 45.000 euros d'amende par ailleurs. J'entends également les critiques souvent caricaturale faites à l'encontre de ce texte sur le droit au logement. je pose notamment l'article 2 de terre qui pérennise un dispositif expérimental issu de la loi Elan luttant simultanément contre les vacances des locaux et contre l'occupation illicite.

contre les cas de squat mais également à mieux prendre en compte les parcours de vie parfois difficiles auxquels sont confrontés certains des locataires de bonne foi et la bonne foi. C'est un des thèmes que je retiens de ce texte. Ici il est pris en compte toutes deux totalement dans ce texte, c'est l'objet du chapitre de de sexe, proposition de loi rassurer les propriétaires sur les risques d'impayés en réduisant les délais de procédure tout en assurant l'accompagnement social des locataires défaillants, sans en faire payer le prix par les propriétaires. Je me réjouis à ce titre de la commune que la Commission rétablisse les pouvoirs de d'du juge. Pour définir le plan d'apurement de la dette locative ainsi que le renforcement des pouvoirs de la CAPEX, ex-commission de coordination des actions de prévention d'expulsion locative au bénéfice d'un meilleur accompagnement social des locataires aujourd'hui nous poursuivons ce travail d'accompagnement des locataires en proposant d'autres modifications supprimer la réduction du délai de deux mois à 6 semaines du commandement afin d'éviter le recours à la procédure judiciaire en permettant au locataire de rembourser la dette. On pourra même sur ce sujet, voir les amendements que nous pourrions voter clarifier le rôle respectif de la CAF et de la CAPEX en cas d'impayé d'un allocataire, mes chers collègues. Nous souhaitons simplement par cette proposition de loi je vous hein. J'habite à en faire de même pour 3 raisons. Première raison sanctionné plusieurs Vermand. Les cas de squat en second lieu, favoriser les traitements à l'amiable des litiges entre propriétaires et locataires défaillants et en 3ème lieu, renforcer la prise en charge sociale de ces mêmes locataires je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame la présidente, Valérie Létard. Pour le groupe Union centriste et pour quatre minutes ne courait pas chers collègues. Madame la présidente. Messieurs les ministres. Madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Le texte que nous étudions aujourd'hui vise à rééquilibrer les rapports locatifs, alourdi par des procédures trop longues et complexes. Et de garantir un renforcement des moyens d'action face à l'occupation illicite des logements. qui nous qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale était endurcis de sanctions qui logé à la même enseigne squatteurs et locataire défaillant. Il était donc avant toute chose primordiale, comme vous l'avez fait. Madame, monsieur le rapporteur de distinguer les squats pour lesquels la législation doit être renforcée des situations d'impayés de loyers souvent liés à des accidents de la vie des locataires et qui requiert un accompagnement précoce et adaptée. À ce type je tiens bien sûr à saluer le travail mené par nos rapporteurs Dominique Estrosi Sassone et André Reichardt qui ont nettement rééquilibré l'organisation du dispositif. La graduation des peines et qui ont su se saisir du sujet complexe des impayés de loyer auquel je m'attache particulièrement dans mon intervention en effet à l'aune des échanges que j'ai eue avec les professionnels de terrain de mon département, j'ai déposé des amendements allant dans le sens de la position défendue par les apports les rapporteurs et qui vise à en préciser ou modifier certains aspects, je vous les expose rapidement tout d'abord, il me paraît nécessaire de rétablir le délai initial de 2 mois entre la délivrance du commandement de payer et l'assignation en justice tous les acteurs de terrain nous le disent. Dans ce laps de temps plus de deux tiers des problèmes d'impayés sont résolus à l'amiable, une réduction du délai mettrait à mal la capacité déjà contrainte des services sociaux à se coordonner et se saisir des situations et ça pourrait générer un effet inverse escompté concernant la procédure contentieuse du litige locatif pour une meilleure réactivité et permettre de rentrer en contact avec la personne concernée par un autre moyen que l'envoi d'un courrier, il apparaît indispensable de communiquer ses coordonnées téléphoniques et adresses mails je propose donc que cette transmission de coordonner soit indiqué dès la rédaction du bail. Afin de préserver un climat de confiance, le partage d'informations doit être le plus lisible possible pour les personnes défaillante. Je propose donc que les informations communiquées par les travailleurs sociaux et médico-sociaux élément strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des ménages au regard de la menace d'expulsion le soir avec l'accord du locataire en respect des règles de déontologie. Enfin s'il apparaît nécessaire de durcir les sanctions s'appliquant à toute occupation frauduleuse d'un logement d'autrui il apparaît tout aussi nécessaire de graduer de de garder le sens de la graduation une peine de prison de 6 mois pour un locataire de défaillant en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement de quitter les lieux. Me paraît. Pas la bonne réponse, ce pourquoi moi je propose de maintenir comme seule sanction les 7500 euros d'amende. Plusieurs aspects méritent aussi notre attention concernant la prévention des impayés de loyers. Elle restera toujours la meilleure politique à privilégier pour éviter les situations trop souvent vécus comme des traumatismes par les familles et comme des injustices par les propriétaires, nous le savons, une part importante des impayés a pour origine le conflit locatif à défaut d'information et de relais à mobiliser les locataires ont souvent comme seul outil défense de leurs droits de locataire, la suspension du versement de loyers, il faut absolument assurer une meilleure identification des acteurs compétents pour agir en faveur de la réduction de ces conflits locatifs relevant de la compétence du réglementaire, cette action se doit d'être renforcée pour mieux prévenir les situations d'impayés concernant le rôle de l'AKP que cela a été répété à plusieurs reprises la coordination des acteurs est essentielle pour agir efficacement dans la prévention des expulsions. Je suis convaincu qu'il faut conforter la cape dans ses actions et en faire le pilier central de cette prévention de l'expulsion tout au long de la procédure. Je salue d'ailleurs le travail de la rapporteure Dominique mais si cher collègue. Toutes mes excuses. Monsieur François Bonhomme. À la parole pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux. Madame, monsieur le rapporteur. La proposition de loi qui nous occupe ce soir vise à mieux protéger les propriétaires de logements contre les squats. Rien de plus. En effet, pour les propriétaires qui découvrent qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux dans leurs propres logements car il occupé illégalement alors même qu'ils sont tenus d'entretenir leurs logements, ils finissent par se retrouver engagés dans une procédure souvent lourde et complexe impliquant des frais d'avocat. Nous avons tous en tête des situations profondément injustes, notamment pour les propriétaires modestes qui ont acquis un logement grâce au fruit d'années de travail. L'actualité récente dans la presse s'est fait largement écho a été ponctuée de situations dramatiques de squat qui ont indigné à juste titre tous les Français. Voilà la raison d'être de ce texte, texte équilibré et je veux saluer ici le travail de notre commission des lois ne rapporteur soucieux d'acc sur et un équilibre entre la nécessité de lutter plus fermement contre les squats et l'indispensable sécurisation des rapports locatifs. Reprenant une partie des travaux déjà menés et qui l'avait conduite à voter en 2021. La proposition de loi de Dominique Estrosi Sassone visant à garantir la propriété immobilière contre le squat. Dont plusieurs dispositions ont été reprises dans le texte de l'Assemblée. En distinguant notamment sur le plan pénal la situation de squatteurs entrés dans des lieux illégalement de celle du locataire qui rencontrent des difficultés pour régler sur le loyer. Pour mieux garantir le droit de propriété. Elle a crée une nouvelle infraction sanctionnant l'eau squat de locaux qui ne constitue pas un domicile élargi au logement qui ne constitue pas un domicile le Champ d'application de la procédure d'évacuation forcée prévu par la loi Dalo. Notre texte. Ne vise donc pas les comportements malhonnêtes. Que les comportements malhonnêtes et non les locataires défaillants, rencontrant une situation économique difficile naturellement. Il est important par l'Allemande d'accompagner au mieux les personnes qui ont du mal à payer leurs loyers, ainsi que de favoriser les conditions. Afin Afin de prévenir une telle situation. Mais c'est précisément parce que des mesures d'accompagnement existe que nous devons également renforcer fortement les moyens de lutter contres les squats. Rappelons que ce droit de propriété est un droit fondamental consacré par l'Assemblée constituante de 1789 dans son article 17 de la déclaration ce droit est un des fondements même de notre société. C'est pour cette raison que le Sénat a souhaité notamment créé la sanction de l'incitation au squat Un service public pénalise la propagande ou la publicité en faveur des méthodes visant à faciliter ou inciter au squat par une amende de 3750 euros. Il est en effet légitime que ceux qui font la publicité pour encourager et faciliter le squat savent à quoi s'en tenir. On a vu ces dernières années fleurir des guides ou des manuels du parfait squatters expliquant avec méthode comment procéder pour préparer son occupation illicite sans risque et s'y maintenir, au mépris des droits du propriétaire. Il s'agit là d'une insulte pour tous ceux qui voient leur droit fondamental de propriété bafoué et nié car ils rompent le pacte social républicain. Plus insidieux ou plus sournois. Quand je vois la Ligue la mal nommée il dit des droits de l'homme alors même que nous avons pris la précaution de distinguer des situations considéré je cite que ce texte vise à criminaliser les victimes de la crise du logement. Ou encore affirmé je cite encore, qu'il s'attaque à toutes les personnes en situation de pauvreté ou de mal-logement il y a là une volonté de trancher les choses et d'ignorer le travail minutieux des du du législateur. Tout cela par pur dogmatisme ou encore la défenseure des droits. Qui n'a aucune considération. Pour les victimes propriétaire et ne s'est nullement à aucun moment. Auto-saisi en leur faveur. Et nous dire que ces mesures n'auront au. Je m'interroge, y aurait-il 2 poids 2 mesures, y a-t-il. Ou plutôt, il y a là une lecture hémiplégique et sélectif dans la défense des intérêts fondamentaux des propriétaires. Parler d'acharnement contre les squatteurs de discrimination ou de criminalisation dans tous les cas, ces propos ces termes sont hors de propos et renvoyé ces situations d'occupation délibéré est caractérisé par des squatters professionnels et se contenter de noyer tout cela sous le prisme de la crise du logement. Je vais voir un déni de réalité. Quand je vois comme minimise la situation de squat, un phénomène marginal, je m'interroge. Oui le contentieux locatif n'a cessé de s'aggraver, dernières années essayer de traiter les cas les plus lourde occupation illicite d'une nécessité pour rétablir la confiance des propriétaires qui se sentent floués. Après avoir vécu ce genre de situation oui nous assumons de renforcer les droits des propriétaires victimes, victimes de procédures interminables. Telle est la raison pour laquelle cette proposition de loi enrichi par le Sénat relève d'une impérieuse nécessité pour établir un début d'équilibre en faveur des propriétaires floués. La parole est à madame Else Joseph. Pour le groupe Les Républicains pour quatre minutes. le monsieur. Messieurs les Ministres mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Si nous examinons ce texte adopté par nos collègues de l'Assemblée nationale, c'est parce que les problèmes subis par les propriétaires, confrontés à des occupations qui n'ont pas voulu persiste. Non le squat n'est pas une opération festive un acte de justice sociale ou une transgression qu'on pourrait comprendre si l'occupation illicite d'un bien immobilier qui porte préjudice aux droits légitimes d'un propriétaire un propriétaire privé des différentes facultés qui constitue classiquement le droit de propriété. Un propriétaire découragé parce qu'il se heurte à des difficultés juridiques et judiciaires, un propriétaire qui enfin doit subir un maquis de procédures et des délais souvent trop long. Le terme peut contribuer à brouiller les consciences par un terme anodin on connoté. Il y a 2 ans, ma collègue Dominique Estrosi Sassone et plusieurs sénateurs avaient déposé et adopté une proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière. Nos collègues députés ont fait le choix de déposer un texte différent mais il reprend des dispositions de notre texte qui mettait le doigt sur des problèmes réels. Je veux saluer cette avancée. Plusieurs points de notre droit pénal mérité d'être. Notre assemblée a été source de propositions. Nous nous réjouissons d'abord de la création d'un délit spécifique d'occupation frauduleuse d'un logement appartenant à un tiers. Il y a aussi l'exécution des décisions de justice leur adoption ne suffit pas à mettre fin à une occupation devenue doublement illicite avec la violation d'une décision du juge. Le maintien son droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire qui a donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de 2 mois sera donc aussi puni. Ces 2 dispositions n'affecte pas les locataires qui bénéficierait de la trêve hivernale ou d'une décision de sursis à expulsion. D'autre clarification sont bienvenues. La peine encourue par l'auteur du délit de violation de domicile et portée à 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, c'est ce que prévoyaient notre proposition de loi sénatoriale. Sur ce point, il fallait aussi clarifier par une peine dissuasive, identique au délit de maintien sans droit ni titre. De même dans cette optique de clarification. Du délit de violation de domicile. Le délit est caractérisée, y compris lorsque le logement a été inoccupés et qu'il contient des meubles, peu importe qu'il constitue ou non la résidence principale de la personne y ayant son domicile. Le délit de violation de domicile est également caractérisé alors même que l'électricité et l'eau était coupée. Ces précisions mette fin aux failles de la jurisprudence actuelle habilement exploitée par des personnes mal intentionnées. Autre dispositif bienvenue. Le constat de cette occupation par des huissiers et par le maire qui devait qui devrait être davantage associés. Mais la lutte contre ces occupations illicites suppose que d'autres comportements soient incriminé ainsi se faire passer pour le propriétaire d'un bien en vue de sa location est aussi est aussi puni comme la publicité en ligne en faveur des méthodes qui visent à faciliter ou incité au squat qui serait punis. C'est également une initiative de notre proposition de loi. Enfin et surtout le propriétaire doit être appuyé ainsi alors qu'il est lésé dans l'exercice de son droit de propriété, il serait paradoxal que la législation n'en tiennent pas compte. Faisant comme si de rien n'était. Le régime de responsabilité de l'occupant sans droit ni titre devrait être. Le propriétaire doit donc être libéré de son obligation d'entretien du fait de l'occupation illicite. Le propriétaire doit être aussi appuyer en amont et pas que pendant l'occupation illicite, le bailleur doit être protégé dans l'exécution du contrat de bail. Le travail du juge ne doit pas seulement s'intéresser à une occupation illicite et à ses conséquences, mais aussi à l'exécution du contrat qui peut être aussi problématique. Ainsi l'inclusion systématique dans le contrat de bail d'une clause de résiliation de plein droit et bienvenue. Mes chers collègues, nous voterons donc pour ce texte avec les amendements approuvés par la commission des lois. Je me réjouis que la voix du Sénat pour aider les Français dans leur vie quotidienne soit écoutée. Merci cher collègue. La discussion. On générale est Close. Nous passons la discussion du texte de la commission. Il y a l'article 1er âge j'ai deux amendements identiques de suppression de 36 Monsieur Merci madame la présidente. Cet amendement est un amendement de suppression de cet article. Par cet amendement. Nous entendons affirmer que les personnes qui n'arrivent plus à payer leurs loyers ne sont pas des délinquants. L'article 1er ah reflète de façon singulière. Les priorités de l'auteur de ce texte. En instaurant un nouveau délit visant à pénaliser l'occupation sans droit ni titre de tout local à usage d'habitation. Il s'agit économique fut une résidence secondaire, un appartement dépourvu de meubles ou un local commercial désaffecté. L'Arctique fait primer de manière absolue la propriété immobilière sur la nécessité pour une personne de disposer d'un logement. Par ailleurs, en visant également les locataires défaillants. Cette disposition fait des personnes ayant du mal à payer leur loyer, de véritables délinquants condamnés des personnes en grande difficulté financière d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 4 fois le RSA est aussi juste qu'absurde. Cela ne les aidera en aucun cas à régulariser leur situation mais aggravera avec certitude leur précarité financière. Notre groupe ça qui a également des nouveaux pouvoirs conférés par cette disposition, aux marchands de sommeil en ce que les locataires titulaires de bail verbal victimes de propriétaires est délicat ou d'un faux bailleur pourraient être pénalement sanctionné. Nous ne cessera de le répéter, au cours de l'examen de ce texte, ce n'est pas par choix, mais bien par nécessité que l'énorme majorité des personnes choisissent de se bâtir dans le logement lors des procédures d'expulsion, notamment en raison de l'absence totale de solutions pour se reloger. Alors que les pouvoirs publics peinent à résoudre la crise du logement et que l'inflation générale des prix aggrave des situations de précarité. merci madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues. À travers cet amendement de suppression et sans reprendre bien évidemment tout ce qui a été dit précédemment, je crois d'abord que nous sommes là effectivement au coeur de ce texte finalement avec 2 projets qui peuvent s'opposer qui peuvent même s'affronter dans le respect du débat démocratique. Tout d'abord, et nous l'avons entendu. Finalement, ce débat est biaisé. Preuve s'il en est d'ailleurs que cette proposition de loi n'est pas à la hauteur des enjeux du moment. Elle vise à opposer. Un droit à la propriété. Et elle avec celui d'droit également fondamental qui est celui de pouvoir se loger pour pouvoir vivre dignement. Oui ou non. La façon dont nous sommes logés a un impact sur les femmes et les hommes que nous sommes, mais plus largement sur les citoyens qui font société ensemble. Nous nous sommes convaincus viscéralement que oui et je le redis, y compris les périodes de confinement que nous venons de traverser l'ont démontré la qualité du logement est indispensable à la qualité de vie. Or, que se passe-t-il aujourd'hui. Les les hébergements d'urgence sont saturés. Le besoin et donc la construction en matière de logements sociaux n'est pas à la hauteur des besoins. Alors j'ai entendu Monsieur le Ministre votre plaidoyer en faveur de ce qui a été fait ces dernières années. Je pourrais vous rétorquer que ce même quinquennat précédent à baisser les APL a fragilisé les bailleurs sociaux dans leur capacité à construire davantage pour mieux répondre aux besoins, mais en tout état de cause in fine et et comme l'a rappelé notre collègue Bernard Roche juste avant sur ce même amendement la réponse que vous faites qui finalement visent à criminaliser celles et ceux qui aujourd'hui sont locataires en difficulté n'est pas à la hauteur des besoins. Merci cher collègue. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur.

Comme vous l'avez vu, la commission a retouché. L'article 1er à pour mieux délimiter le Champ des infractions et instaurer une meilleure gradation dans l'échelle des peines. Mais elle ne souhaite pas pour autant. Supprimer entièrement cet article, considérant qu'il est important de garantir le respect du droit de la propriété aujourd'hui le code pénal sanctionne seulement le squat du domicile au nom du respect de la vie privée, ce qui ne nous paraît pas suffisant pour couvrir toutes les situations. Je vous remercie. Mais c'est l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. ce que vient de dire monsieur le rapporteur est parfaitement juste. Nous sommes dans une situation aujourd'hui qui ne couvre pas. Toutes les réalités. D'où la nécessité de légiférer, pas pour le plaisir. Alors je voudrais quand même dire. À Madame. La sénatrice qui. Monsieur le Sénateur, mélange de choses. Criminalisé. Criminaliser les pauvres au au fond c'est ça. Vous ne le dites pas mais c'est présent dans votre esprit. Ce sont des mots qui sont excessifs je veux dire pourquoi. Le procureur. Ah toujours la possibilité d'un classement sous condition. Conditions de partir par exemple. Le tribunal pourrait retenir dans certains cas extrêmes, l'état de nécessité. Quant à l'amende. Monsieur sénateur mais arrange vous dites. 30.000 euros d'amende soit X fois le SMIC. Mais vous savez que un prévenu quand il comparaît devant la juridiction pénale. On lui demande systématiquement d'amener des justificatifs de revenus parce que le juge a l'obligation. Lorsqu'il envisage de prononcer une amende de la moduler en fonction des facultés contributives. De sorte que ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. Tout à fait exact. Bon on va sortir de ces postures idéologiques. On a envie je crois personne d'entre nous de criminaliser ce qu'on veut c'est que. Oui on couvre toutes les situations qui sont celles de notre actualité de notre réalité et qu'on ne puisse plus tout simplement squatter des locaux quand ils ne vous appartiennent pas. Voilà les choses me semble plus juste. Dans cet ordre là. Donc madame la présidente. Je suis défavorable à ces amendements. Merci monsieur le ministre alors je mets aux voix Madame Lienemann. Je ne veux pas parler d'idéologie encore que ce mot ne soit pas un gros mot. Parce que je crois que c'est quand même important qu'. On est certain, les uns les autres, une certaine lecture de comment on imagine la République. 1er point les locataires qui n'ont pas pu pays. Si le gouvernement considéré cette sur ce sujet à nouveau comme très important même si les chiffres sont à dire que jusqu'à ce jour. Croisons les doigts. Il y a pas eu d'augmentation. Il aurait dû consulter. Consulter les acteurs consulter élus locaux. Reprend le débat sur la garantie universelle des loyers qui je le rappelle. A été votée par les 2 assemblées. Avec nos collègues Mézard dont chacun sait que c'est quand même pas bolchévique. Qui avait été le rapporteur de cette solution. Qui ne crie n'est pas le pays.

Elle avait l'immense Avantage. D'obliger les propriétaires qui voulant en bénéficier. De signaler dès le 2ème mois d'ailleurs Dominique reprend cette thèse du mois auprès des comités pour voir si la personne avait besoin d'aide sociale ou si elles étaient potentiellement de mauvaise foi. Mais dans tous les cas de figure, le propriétaire était payé. Et la se retourner contre et propre. Les locataires de mauvaise foi. On aurait pu reprendre ce débat.

Merci madame la présidente n'entrer très rapidement parce que j'ai, j'ai l'impression que là sur ce sur ce texte on part c'est comme si on partait de rien mais il me semble et d'ailleurs Monsieur le Ministre de la rappeler que la violation de domicile. C'est pour l'instant un an de prison et 15.000 euros d'amende.

puisque vous même tout à l'heure Monsieur le Ministre, vous l'avez très bien expliqué. En fait c'est la, c'est la question de l'application de des de la peine. Et que voilà, vous aviez une difficulté, donc je pense que là pour le coup il y a une vraie responsabilité sur le comment on peut appliquer ces peines et puis la vraie question, parce que oui c'est bien une une criminalisation de la, de la précarité à travers, à travers ce texte, c'est que oui il y a une question de relogement et la question de ce relogement. Pour l'instant on est dans l'incapacité parce que on n'a pas de politique de logement qui soit satisfaisante et donc c'est bien là encore une fois le problème. Merci alors je mets aux voix donc ces deux amendements qui ont reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ne sont pas adopté

3% des propriétaires possède 50% du parc immobilier locatif. Ont travailler. Juste un petit point de repère, voilà. Moi je voulais vous poser une question. Aux auteurs de la loi je verrai après dans les explications de vote, mais je voudrais que vous nous expliquez bien pourquoi vous avez rajouté. Les logements. Locaux économique. Voilà, je voudrais savoir pourquoi vous avez rajouté les locaux économique. Et comme j'ai pas envie de voir le le mal ou le loup se cacher derrière. Puisque de souvent. On est en plein mouvement social il y a des mouvements sociaux qui font qu'on occupe. À un moment donné, les salariés occupent un lieu. Une activité et caetera. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'est-ce qui vous amène à partir de quelle réalité d'une ampleur considérable. Il y a un problème du point de vue des locaux économique qu'est-ce qui se passe, ce qui nous a échappé du point de vue des squats. Dans les locaux économique qui serait d'une importance telle qu'il faudrait vraiment légiférer ce soir, voilà c'est une demande d'explication et après on verra. Suivant l'explication Merci l'amendement 15 hein. Monsieur le Président Patriat. Je vais très bref dans la présidente l'amendement que nous proposons modifie la notion de local à usage économique. Par la notion de locaux à usage commercial agricole aux professionnels qui sont des notions déjà connu de notre droit. Le Sénat avait d'ailleurs proposé les mêmes termes de la loi de sécurité globale. Par l'ajout du terme, exploiter l'amendement permet également d'exclure du Champ de la répression. L'introduction et le maintien dans des locaux vides et désaffectés par certaines associations du droit au logement. Je vous remercie. Ce sera un avis défavorable sur les deux amendements pour des raisons naturellement différentes s'agissant des différents amendements sur le 61. Cet amendement. Je Savoldelli vise à exclure les locaux à usage économique du Champ d'application de l'article premier. Qui concernerait dès lors les seuls locaux d'habitation. Cette exclusion ne nous paraît pas justifié et je réponds à votre question un artisan, un commerçant un petit chef d'entreprise pouvons voir ses locaux squattés et d'alors son activité économique entravé. Il n'a donc pas anormal à notre avis, que la loi puisse protéger également les locaux à usage professionnel ou commercial contre le squat.

Pour punir l'occupation sans droit ni titre d'un local à usage d'habitation ou à usage économique. Votre amendement Monsieur Patriat propose de remplacer la notion de local à usage économique par la notion de local à usage commercial professionnel ou agricole est ça j'ai pas, pour nous au niveau de la commission d'un simple changement sémantique l'ajout du terme exploiter implique que l'infraction ne serait pas constituer si l'occupation sans droit ni titre concernait un local inexploité. On peut en effet se demander s'il est bien opportun de pénaliser l'occupation par des personnes à la rue de locaux occupations de locaux désaffectés. Toutefois, je vous rappelle que l'objectif du nouvel article 315 tirer 1 du code pénal et de protéger la propriété en privé en tant que tels que le juge À usage économique soient exploités ou non. Prenons garde à ne pas donner l'impression que l'on tolérerait certaines formes de squat lorsqu'elles concernent des locaux inoccupés. D'ailleurs un entrepôt un commerce peuvent être inoccupée pendant une période donnée. Cela ne veut toujours pas dire que le propriétaire n'a pas un projet pour l'avenir. Projet que ce squat pourrait entraver la raison pour laquelle je donne un avis défavorable tant au 1er qu'au 2ème amende. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. merci madame. La présidente, monsieur le sénateur. Ça veut lits vous poser une question, avez-vous dit à l'auteur. Moi je ne suis pas l'auteur. Je rappelle que c'est une PPL. Et Kasbarian. Le gouvernement sur. Cette question avait émis un avis de sagesse. Mais des débats parlementaires, si je puis me faire le porte-, parole de ce que j'en ai compris évidemment. Avec. La subjectivité qui est la mienne. Il s'agissait effectivement comme l'a dit monsieur le rapporteur. De d'envisager les cas où. On viendrait ça s'introduire dans une, dans dans une boutique dans une échoppe. Dans une boulangerie dans je peux voilà et que naturellement il fallait aussi protéger les artisans, les petits commerçants et que ça avait du sens. S'agissant de de de l'amendement déposé par Monsieur le le sénateur. Patriat le gouvernement il y est favorable. Pour. Plusieurs raisons d'abord d'abord pardon parce que. La notion de de local économique ça je pense qu'on en met tous d'accord est une notion qui en droit n'a aucune résonance donc il convient d'affiner les choses. Alors Monsieur le Sénateur Patria propose de retenir local à usage commercial agricole professionnel exploiter. Je rappelle que, à l'origine, nous sommes sur le logement. Et moi, pardon, je fais la différence entre. Un terrain. Grillagé. Et un domicile et une habitation et je ne souhaite pas qu'on les mette au même niveau. Et je pense que la nuance qui est introduite par monsieur le sénateur. Patriat. Doit attirer notre attention. Les choses ne sont pas dans la même gradation dans la même gravité. Nous avons d'ailleurs pour justifier de ce texte à venir pris un certain nombre d'exemples médiatique que nous avons tous vu qui nous on touche beaucoup ému au fond. Et pardon mais là j'imagine mal le propriétaire du terrain dans mon, dans sa caravane et se disant mais je ne veux pas rentrer sur mon terrain. On n'est pas sûr de la violation du domicile avec tout ce que ça comporte. D'effraction dans l'intimité de pénétration dans un logement qui est le logement de sa propre famille. C'est pas la même dimension. C'est la raison pour laquelle moi je souligne la nuance du sénateur Patriat et je souhaite que nous le fassions nôtre. Merci Madame Lienemann. Je désapprouve cet article mais je voterai l'amendement de Monsieur Patriat. Parce que j'ai expliqué pourquoi. Jusqu'à présent. Les gouvernements successifs. N'ont pas voulu sanctionner systématiquement tous les. Tous les squats. Même si on est bien d'accord, on parle plus du domicile occupé qui sanctionnant. C'est que depuis la Libération. Et la le droit à la propriété. A été comparée. À l'intérêt général. Au regard de la crise du logement. À la Libération. On a créé le principe de réquisition. De logements vides ou de locaux vides. Permettant de loger des gens qui n'étaient pas logées. Et le droit à la propriété a toujours été compensé par rapport au droit à l'intérêt général et à l'ordre public. Et comme ce droit là. La plupart du temps l'État ou les collectivités. Ne veulent pas le faire prévaloir, ce qui d'ailleurs est une erreur parce qu'on on paye, on paye le propriétaire. Tandis qu'à squatter touche rien du tout. Comme personne n'a voulu faire ça. Parce qu'évidemment ça coûte. Et bon on a laissé faire du squat. Dans des locaux vides. Logement ou. Le prof, usines désaffectées, etc. La plupart du temps. Ça pose plus de problèmes de cohabitation avec les voisins. Qu'un problème de. Propriétaires. Et donc personnellement, je trouve. Que la la pénalisation supplémentaire dans ce cas-là. Et va faire ressortir des tas de problèmes qui ne seront jamais résolu comme je vous le disais, il y aura pas d'offre. A minima. J'estime que la proposition de Monsieur Patriat, si je puis dire, limite la casse. Et pour ma part et je l'avoue. Merci, cher collègue, Oui je trouve ce débat très intéressant parce que. Le rapporteur nous a bien expliqué qu'en fait. S'il voulait mettre sous la même enseigne en amalgamant la totalité des locaux d'habitation. De. Meubler les locaux commerciaux, les locaux économique. Les terrains les friches industrielles et cetera c'était parce que ce qui prime et d'une manière claire et absolue c'était le droit à la propriété, ils on a bien compris, c'est bien ce qu'on reproche d'ailleurs à ce texte, c'est cet amalgame constant au nom de la propriété de absolue immobilière qui primerait sur tout le reste et c'est bien cela qui fait que nous avons une position et négatives sur ce texte. Le ministre aussi. Je suis totalement d'accord avec sa démonstration a bien montré aujourd'hui qu'il y avait des possibilités de locaux ou de terrains qui n'étaient pas exploitées depuis des années et qui pour les réseaux qu'a expliqué Barid Walid Bad étaient utilisés aujourd'hui pour loger des gens aux dans de l'intérêt public ou aux dents de la capacité de l'État et de l'administration à leur fournir des logements décents. Dans ce cadre-là, nous voterons bien entendu les 2 amendements et nous voterons celui de Monsieur Patriat, parce qu'effectivement pu dire aggraver la pénalisation. Dans le cas de squat sur des. Sur des terrains ou des locaux dans d'exploiter depuis des années et puis dire, de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende le fait pour une association oeuvrant pour le droit au logement qui ne cause aucun trouble alors public d'occuper des locaux vides et exploiter nous paraît absolument inadaptés donc nous votre les 2 amendements.

d'abord qu'il s'agisse de locaux à usage d'habitation de locaux à usage économique que je sache, il s'agit bien d'une propriété privée et donc je ne vois pas pourquoi on excuserait plus facilement une occupation illégale de locaux à usage professionnel qu'une occupation illégale de locaux à usage d'habitation. Je rappelle également que si l'on veut donner toute sa force au dispositif qui est celui du logement intérimaire qui permet à des sociétés privées qui sont agréés par l'État ou à des associations de pouvoir permettre à des gens d'occuper temporairement des locaux qui sont vacants et qui, généralement, ce peuvent être des locaux de bureaux des locaux à usage professionnel pour leur permettent justement le temps de la convention d'occupation de pouvoir être logés. En contrepartie de quoi les sociétés doivent bien sûr entretenir ces 10 locaux c'est aussi pour donner toute sa force à ce dispositif que nous avons voulu pérenniser et qui véritablement apporte des réponses, on l'a dit en terme de logement de personnes en mobilité géographique en mobilité professionnelle. Également de personnes en situation de fragilité. Donc moi je mets vraiment sur le même niveau les locaux à usage d'habitation et les locaux à usage professionnel et je n'excuse l'occupation illégale, ni des uns ni des autres. Merci madame voyez pour une intervention très courte. Madame la présidente. Je souscris tout à fait ce que vient de dire. Madame Estrosi Sassone. Mais permettez-moi d'être surprise. Monsieur le Ministre, vous avez dit sagesse. Mais en quoi est-il sage de dire en fait d'une certaine manière, que ces. Locaux sont squat table. Parce que c'est, ah ça c'est ça que ça veut dire si, s'ils sont si le propriétaire est moins propriétaire et qu'on peut les occuper premièrement et deuxièmement. Ses locaux ils sont peut-être inoccupé, mais les propriétaires de ces locaux, ils payent des taxes ils les entretiennent, ils payent des assurances. Pourquoi leurs biens seraient-ils moins protégés par la loi que les autres en vertu de quoi c'est pas comme si on avait pas de loi sur le logement, c'est pas comme si nous nous étions dans un pays. Sans effort pour les personnes qui rencontrent des difficultés pour le logement. Donc moi j'avoue que je ne comprends pas. L'amendement que je ne voterai pas de de Monsieur Patriat à ce niveau-là parce que je pense qu'il. Non seulement je je suis pas d'accord sur son esprit mais en plus je pense qu'il encourage un trouble. Qui est déjà très important et que nous essayons de combattre dans ce texte sur les occupations illicites et je pense que c'est vraiment un, un encouragement. En tout cas une permission. Vers. Des violations de la propriété qui doivent rester des violations de la propriété, il y a pas des sous, propriété de sur propriété sinon je crois que le Fisc. Hormis des catégories sur les logements quoi les logements Pasqua table mais les propriétaires qui sont victimes de spoliations parce qu'ils sont squattés continue, malheureusement pour eux à payer les taxes, les assurances et cetera et être responsable de leur logement. Monsieur Savoldelli. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues. La la réponse sur le pourquoi des locaux économique je pense être. Le mot locaux économique est pas satisfaisant.

et peut être en vigueur des des processus d'expulsion sans jugement du domicile occupées illicitement. C'est vrai pour les locaux professionnels il y a pas une spécificité à. Trouver. Et deuxièmement, je vous avoue que. Mais là je pense ça mérite d'être vraiment et. C'est que vous comprenez bien qu'il peut y avoir chez des salariés. Qui ne sont pas propriétaires de l'activité économique ni actionnaire de l'activité économique. Le besoin d'être rassurés sur le fait qu'il puisse exercer ce qui est dans le code du travail. Vous voyez quand même faut quand même qu'on qu'on se préoccupe de cette question là quand on aborde le le sujet qui nous est présentée. S'agissant de la l'amendement de Monsieur Patriat. Notre groupe, nous on est pour. Le voter. Qu'il soit discuté dans la navette. Parce que franchement qu'est ce qu'il dit faut pas lui en faire dire plus que ce qu'il ne dit.-il exclu du Champ de l'arrêt, la répression, l'introduction du maintien dans les locaux vides et désaffectés. Voilà donc. Évidemment, on le sait tous nommés. On a tous connu il y a des locaux vides et désaffectés où le propriétaire a des dettes ou le propriétaire ne payent pas d'assurance ou le propriétaire fait des fois des deal pour des raves parties ou autre chose. Nous vous voyez si on prend tous les cas particuliers. On va pas faire loi donc voilà moi je vous dis nous on votera parce que je pense que c'est. C'est un c'est un amendement moins 10 ans. Mais au moins il a le mérite d'ouvrir une certaine À à l'utilisation de locaux qui sont sont surtout vides et désaffectés. Je ne vois pas en quoi c'est l'intérêt de l'économie et du professionnel d'avoir pendant longtemps des locaux vides et désaffectés, autant en avoir un usage qu'ils soient associatifs ou d'autres intérêt c'est sûr. Collègue monsieur le rapporteur. Richard.

et s'agissant de de. Vous avez bien compris que le terme exploiter pose problème par contre Monsieur Patriat vous auriez simplement parlé du substituer le terme à usage économique par commercial agricole ou professionnel, nous aurions naturellement donné un avis favorable puisque ces termes figure bien d'ores et déjà. Dans notre législation mais nous aurons l'occasion de corriger ça dans la navette. Merci, monsieur le Ministre. D'abord, merci madame la présidente. Répondent d'abord à Madame la sénatrice Boyer qui m'interpelle, j'espère que vous ne regrettez pas notre moment de. De communion. Bref, il est vrai, mais qui existe et vous l'avez souligné la sagesse madame la sénatrice, n'est pas la sagesse auto-proclamé du ministre. Quand le ministre dit sagesse. Ça signifie qu'il s'en rapporte à la sagesse des parlementaires. Ce n'est pas de la mienne, dont il est question, non de me demandez pas à moi en quoi il serait sage, je n'ai pas prétendu à la sagesse j'Aspire à la vôtre c'est singulièrement différent pour, pour le reste. Moi je fais la différence enfin pardon bien sûr que tout est interdit, mais on peut t'interdire sans. Texte. Répressif sans texte pénal. Moi je fais le distinguo entre le logement. Un garage exploités et un garage inexploité. D'abord, ça n'est pas Madame la députée. Estrosi Sassone entre un, un logement et et un local. Non plus économique, mais qui seraient exploités artisanale par exemple non ces logements local artisanal exploités. Et lequel inexploité. Ces trois pas de.

Le mot qu'on a utilisé le plus tout à l'heure enfin depuis le début de ces débats. C'est le mot équilibre. Et moi je dis que votre commission a apporté un certain nombre d'enrichissement au texte véritablement. Veillons à ce que on ne regarde pas ce texte en disant on criminalise les pauvres et cetera parce que ça. C'est naturellement totalement. À des années lumière de ce que nous voulons faire, nous voulons rétablir une certaine forme de de justice et point n'est besoin de de. De, de, de crier au loup, si j'ose dire parce que ça n'est franchement pas dans nos intentions. Voilà moi je distingue. On a donné des tas d'exemples tout à l'heure qui nous ont émus. Ben je sais pas moi si la présence d'une famille dans un hangar ça suscite autant d'émotion et donc est-ce que ça peut nous amener vers une décision. De judiciarisation de pénalisation moi je je pense que non et c'est ce que. En appelant votre sagesse, j'ai, j'ai essayé d'exprimer. Merci, monsieur le Ministre, alors je mets aux voix l'amendement 61 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 15 avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté. Alors, mes chers collègues. Je vais lever la séance. Je vous rappelle que la suite de l'examen de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite est inscrite à l'ordre du jour de ce jeudi 2 février 2023 à l'issue de l'espace réservé au groupe geste et éventuellement le soir. La prochaine séance mercredi 1er février 2023 à 14h 30 pour l'allocution de monsieur Rouslan Stefantchouk. Président de la Rada d'Ukraine. La séance de questions d'actualité au gouvernement débutera exceptionnellement à 15h 15, la séance est levée.